Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la lecture d'une déclaration de politique générale du Gouvernement. Je donne la parole à M. François de Rugy, ministre d'État,

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais donner lecture du discours de politique générale, que le Premier ministre prononce en ce moment même à l'Assemblée nationale. Je veux vous dire l'honneur et la fierté que je ressens d'être ici, au Sénat, pour prononcer devant vous ce discours de politique générale. Le fait que je lise mot pour mot le texte du Premier ministre prêtera peut-être parfois à sourire, mais je crois que nous sommes toutes et tous attachés aux règles de notre Constitution. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà deux ans maintenant que nous gouvernons, et il y a toujours urgence- peut-être davantage encore. « Urgence économique, comme le crient les salariés des usines de Belfort, d'Amiens et d'ailleurs. « Urgence sociale, comme le crient nos concitoyens des territoires isolés, comme le disent les personnels hospitaliers. Urgence écologique, comme le crient les jeunes Français à l'encontre des gouvernements et des entreprises qui n'en font pas assez. « Urgence politique : le 26 mai, l'extrême droite est arrivée en tête des suffrages en France. » Ce n'est pas un hasard ! « Comme dans beaucoup de démocraties occidentales, la radicalité politique, nourrie de l'obsession du déclin et de la peur de l'autre, structure désormais une part de notre vie démocratique. Cette urgence, elle nous rassemble : c'est elle qui a conduit à l'élection du Président de la République ; c'est elle qui a donné une majorité au Président de la République lors des élections législatives c'est elle encore qui a guidé votre vote de confiance au Gouvernement il y a deux ans, pour conduire un intense agenda de transformations. Je ne reviendrai pas ici sur la longue liste des réformes que nous avons menées les Français n'attendent pas un bilan, encore moins un exercice d'autosatisfaction. Je veux simplement dire au Gouvernement et à la majorité que j'en suis fier et que je les remercie du travail accompli. Le chômage est au plus bas depuis dix ans, l'investissement au plus haut depuis douze ans, la progression du pouvoir d'achat la plus dynamique depuis dix ans

Nous n'avons eu de cesse, ces deux années durant, de tenir le cap fixé par le Président de la République. Celui que nous jugions nécessaire pour libérer les forces de notre pays et protéger ses citoyens, quitte à prendre des décisions impopulaires, quitte à commettre des erreurs, et j'en prends évidemment ma juste part. Quelles qu'aient été les difficultés, l'essentiel des mesures annoncées dans ma précédente déclaration de politique générale est aujourd'hui engagé. Cette fidélité à la parole donnée a forgé la légitimité de notre action. « En novembre dernier, nous avons rencontré la colère. Certains diront que nous l'avons seuls créée. Je ne le crois pas. Cette colère vient de loin, et bien des démocraties l'ont ressentie dans des formes variées. Mais peu importe. C'est à nous, gouvernants, parlementaires, qu'elle était en premier adressée. D'une certaine façon, elle nous rappelait à notre promesse de promouvoir le travail et de lutter contre les injustices. Nous avons décidé des mesures puissantes pour répondre aux aspirations des Français et pour apaiser. « De cette période, qui m'aura marqué profondément- comme, je crois, chacun d'entre vous vous -, puis du grand débat, qui a permis à des centaines de milliers de Français de se rendre dans leur mairie ou dans des salles publiques pour dialoguer, travailler et réfléchir, le Gouvernement et la majorité entendent tirer la force d'un nouvel élan. C'est " l'acte II " du quinquennat ; une nouvelle étape qui marque une césure, à travers un profond changement de méthode, mais qui va de pair avec deux impératifs : la constance et la cohérence, qui sont bien les seules choses que notre pays n'ait jamais tentées. « Constance et cohérence dans l'action. Notre pays a besoin de se transformer. Notre ennemi, ce n'est pas le mouvement, c'est le. « Constance et cohérence dans nos valeurs ensuite. Nos valeurs, ce sont le patriotisme, l'attachement à la République, l'affirmation de l'idéal européen. C'est la quête de justice sociale, pas celle qui se paye de mots, mais celle qui se vit au quotidien. C'est la valeur travail, cette idée simple que les solutions proviendront du travail et qu'il faut donc le récompenser. C'est le dépassement des postures et des vieux clivages. Plus que jamais, notre pays a besoin de l'union des Françaises et des Français qui veulent agir, loin, bien loin, des logiques partisanes. L'engagement partisan est évidemment respectable.

prévoie qu'ils concourent à l'expression du suffrage universel. Les partis demeurent donc des acteurs centraux de la démocratie. « Je ne crois pas, pour ma part, que les cultures de gauche et de droite aient disparu.

Mais ces cultures suffisent-elles à structurer le débat ? Disent-elles quoi faire sur l'Europe, sur l'écologie, sur la politique méditerranéenne, sur la décentralisation ? Je ne crois pas, mesdames, messieurs les sénateurs, que le vrai sujet soit aujourd'hui de savoir comment ressusciter la gauche ou sauver la droite. Le but est de savoir comment, avec nos héritages, nos sensibilités, nos différences, nous dépassons nos habitudes, pour nous rassembler, pour relever les défis de notre pays et de notre planète.

Car nous avons beaucoup fait depuis deux ans, mais il reste tant à faire ! « Au coeur de l'acte II, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela, le dépassement des anciens clivages. « Je connais les soupçons me concernant »- c'est le Premier ministre qui parle ! Je Je répète fidèlement ce que dit le Premier ministre à l'Assemblée nationale en ce moment. « Je viens de la droite, j'ai travaillé dans une grande entreprise française du nucléaire, je suis élu d'une ville industrielle, je ne pourrais donc ni rien comprendre ni rien faire. » C'est évidemment toujours le Premier ministre qui parle, mais sachez que, moi qui ai une histoire différente, un parcours différent, je suis fier de servir sous ses ordres et ceux du Président de la République. Je trouve que c'est faire peu de cas de ma culture politique, de mon expérience au Havre »- pour ma part, je pourrais dire à Nantes -« et de ces deux années de gouvernement. Mais oui, j'ai mis du temps, comme d'autres Français, à considérer que ces enjeux étaient aussi urgents que la défense de l'emploi ou la sécurité. Les jeunes nous bousculent, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité. « Je ne me ferai pas passer pour un autre : je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois dans la science. » Très bien ! « Je voudrais qu'elle ait plus de place dans le débat public, que nos décisions soient davantage éclairées par elle. Je sais ce que notre pays doit à son agriculture et la chance qu'il a de pouvoir compter sur des agriculteurs exigeants et passionnés. J'aime l'industrie : j'admire ses salariés, ouvriers, techniciens et ingénieurs. Je crois en l'économie de marché régulée par le politique, en l'innovation et en la force de la croissance. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. Et je crois qu'à chaque fois que nous mettons une incitation financière publique en place, il faut s'interroger sur son efficacité réelle ... C'est vrai ! ... et songer à la façon dont les acteurs privés prendront un jour le relais. Il faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction, et je veux être jugé sur les actes. Car ces douze prochains mois seront ceux de l'accélération écologique. » Bravo ! « Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie, et tout d'abord notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des deux projets de loi dont vous êtes saisis

C'est ce gouvernement qui fermera la centrale de Fessenheim, avant la fin 2020, et qui a proposé un chemin crédible pour réduire la part du nucléaire à 50 % d'ici à 2035, avec le développement massif du renouvelable et notamment de l'éolien en mer. En arrivant aux responsabilités, nous avons concrétisé et considérablement baissé les coûts de six appels d'offres qui étaient bien mal partis. Aujourd'hui, le projet au large de Dunkerque démontre que les coûts baissent encore plus vite quand les projets sont bien montés. Nous pourrons ainsi augmenter le rythme des futurs appels d'offres à un gigawatt par an.

à Gardanne, Saint-Avold, Cordemais, Le Havre, où les centrales à charbon fermeront d'ici 2022. « Le succès de la prime à la conversion pour l'achat d'un véhicule moins polluant nous permet de doubler notre objectif : nous visons désormais 1 million de familles d'ici la fin du quinquennat. « Nous donnerons une nouvelle orientation à notre politique hydroélectrique. En la matière, on ne régule pas seulement une production électrique, mais des vallées et des régions entières. Nous respecterons le droit européen, mais nous n'accepterons pas le morcellement de ce patrimoine commun des Français. Enfin, nous négocierons avec la Commission européenne une nouvelle régulation du prix de l'électricité, pour que les Français bénéficient davantage de la stabilité et de la compétitivité que nous donnent nos investissements passés. Nous voulons donner aux Français les moyens de se chauffer sans polluer ni payer toujours plus. « Nous remettrons totalement à plat les aides existantes à la rénovation énergétique, parce que ces aides sont d'une effroyable complexité, qu'elles profitent en réalité aux ménages les plus riches. Nous transformerons donc le crédit d'impôt de transition énergétique en une aide plus massive, versée en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Reconnaissons-le, à part dans le logement social, nous ne disposons pas aujourd'hui des leviers efficaces pour venir à bout des passoires thermiques qui plombent le climat et le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Inventons-les ensemble ! Je sais que les parlementaires

raisonner au-delà des normes et des obligations, même si elles sont nécessaires, et réitérer le succès qu'un Jean-Louis Borloo a pu avoir avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine en son temps. Le deuxième axe de notre plan de bataille, c'est de rompre avec le gaspillage, d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. « J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu »- alors que c'est encore neuf. « Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage, qui sera l'une des trois priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Nous avons déjà acté la suppression des produits plastiques à usage unique les plus néfastes. Mais je veux que nous allions plus loin. « Parce que l'État se doit d'être exemplaire, tous les produits en plastique jetables seront bannis de l'administration à compter de l'année prochaine. Je souhaite également que nous nous fixions un objectif de 100 % de plastique recyclé, et nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation, notamment avec les collectivités locales, pour étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. Les collectivités d'outre-mer pourront, si elles le souhaitent, en devenir les territoires pilotes. La loi anti-gaspillage prévoira la possibilité d'imposer l'incorporation de plastique recyclé dans toutes les bouteilles en plastique à usage unique. j'ai noté la volonté de beaucoup de parlementaires d'aller plus loin dans la suppression du plastique à usage unique. Un amendement avait étendu cette obligation à toutes les boîtes plastiques. Nous avions considéré ensemble qu'il ensemble qu'il déstabilisait trop nos industries et qu'il fallait le corriger. Mais son intention était bonne, et je vous proposerai dans le cadre de la loi anti-gaspillage des dispositions pour interdire progressivement les boîtes plastiques qui ne sont pas constituées de plastique recyclé. S'agissant de l'alimentation, nous devons produire et manger mieux. « Nous nous battrons en Europe- le Président de la République l'a réaffirmé -pour garantir un budget de la PAC à la hauteur des besoins de la transition écologique, un budget qui protège nos agriculteurs et qui leur donne les moyens de produire autrement. Nous réorganiserons également notre police de l'alimentation pour apporter aux Français davantage de garanties sur ce qu'ils consomment. « Nous avons Nous avons lancé avec succès une démarche nationale pour améliorer l'information sur la qualité nutritionnelle des aliments et développer l'utilisation de nutri-score dans l'étiquetage des aliments. Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires, afin de rendre le nutri-score obligatoire. « Un mot pour conclure sur ce point : en matière de prévention, le Gouvernement a un bilan que je crois solide, sur le tabac, les vaccinations, la sécurité routière. Agnès Buzyn m'a proposé d'ouvrir une nouvelle étape, pour s'attaquer à l'obésité. Il s'agira d'un objectif national, pour l'école, la santé, le sport, l'agriculture, l'industrie. Je serai heureux d'accueillir les propositions parlementaires sur ce sujet. personne -« je souhaite que les Français soient les premiers acteurs de la transition écologique. La convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le Gouvernement s'engage à traduire ces propositions en projets de loi, en mesures réglementaires, voire, pour les plus puissantes, à les soumettre à référendum. Le conseil de défense écologique s'assurera, pour sa part, de la mobilisation au plus haut sommet de l'État pour faire de l'écologie une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques. Nous devons défendre aussi bien le climat que le pouvoir d'achat, la qualité de l'air que nos industries ou nos emplois. Nous avons là un nouvel " en même temps " à construire, qui appelle les mêmes dépassements : dépassement des oppositions entre producteurs et écologistes, dépassement de nos habitudes de consommation, dépassement des postures. Il faut que nous arrivions à en faire l'affaire de tous. Et il faut que nous nous concentrions sur les résultats concrets, dans le quotidien des Français. Je ne veux pas être l'homme des effets d'annonce, mais celui des engagements tenus.

Le chômage baisse ; il a même atteint son plus bas niveau depuis dix ans. Avec 93 000 emplois créés au premier trimestre, les chiffres publiés encore ce matin par l'Insee montrent que nous sommes sur la bonne voie. nous n'en avons pas fini avec un chômage de masse qui enferme dans la précarité, qui lamine des familles et des territoires. Chaque période de chômage est une épreuve, est une angoisse. C'est un combat de tous les jours pour celui qui y est confronté. C'est le combat central de mon gouvernement, car nous en avons fini avec la résignation et l'idée délétère que tout aurait été tenté contre lui. Nous avons renforcé le dialogue social dans l'entreprise, pour mettre fin à la peur de l'embauche. Nous avons réformé la formation professionnelle et l'apprentissage, pour développer les bonnes compétences en face des besoins. Nous avons mis en place un plan Pauvreté dont l'objectif central est la reprise d'activité. Il faut maintenant achever ce vaste mouvement de réformes et conduire, comme tous nos voisins l'ont fait, celle de notre assurance chômage. « Avec la ministre du travail, Muriel Pénicaud, nous présenterons la réforme mardi prochain, le 18 juin. Nous nous fixons plusieurs objectifs. Le premier, c'est de mettre fin au recours abusif aux contrats courts. « Nous avons donné aux entreprises plus de souplesse et de sécurité grâce à la réforme du droit du travail, et c'était nécessaire. La contrepartie- vous savez combien j'apprécie ce terme -, c'est une responsabilité accrue dans le recours aux contrats courts, qui empêchent les salariés de construire leur vie avec un minimum de sérénité. C'est pourquoi, dans les cinq à dix secteurs d'activité qui utilisent le plus ces contrats et qui génèrent de la précarité, nous instaurerons un principe de bonus-malus sur les cotisations d'assurance chômage. Dans les autres secteurs, nous prendrons une mesure transversale pour décourager le recours aux CDD d'usage. « Le deuxième objectif de cette réforme, c'est de faire en sorte que le travail paye toujours plus que l'inactivité. C'est en général le cas. Dans la majorité des situations, les règles d'indemnisation sont bien faites et elles continueront à s'appliquer. il existe des situations où le montant de l'allocation mensuelle du chômage est supérieur au salaire mensuel moyen perçu. Nous devons y mettre fin. Le troisième objectif vise à introduire une dégressivité de l'indemnisation pour les salariés qui perçoivent les salaires les plus élevés et qui sont en mesure de retrouver un emploi plus vite que les autres. Quatrième objectif de la réforme de l'assurance chômage : renforcer l'accompagnement des demandeurs d'emploi. « Vous le savez, le Gouvernement a regretté que les partenaires sociaux n'aient pu, par le dialogue, réformer eux-mêmes le régime d'assurance chômage, mais nous continuons à penser qu'ils ont leur place dans la mise en oeuvre de cette réforme, comme ils ont leur place dans la mise en oeuvre de tout l'acte II. En particulier, En particulier, les nouvelles mesures d'accompagnement, pour lesquelles nous dégagerons de nouveaux moyens, ne doivent pas être pensées uniquement à Paris : les besoins ne sont pas les mêmes selon les bassins de vie et d'emploi. Les travaux que j'ai lancés autour de la mobilisation nationale et territoriale avec les partenaires sociaux »- et les élus locaux -« devront permettre d'identifier les meilleures solutions et donner une grande marge de manoeuvre aux acteurs locaux. J'ajoute que, conformément aux engagements du Président de la République, cette réforme donnera accès à l'assurance chômage aux salariés démissionnaires, ainsi qu'aux travailleurs indépendants. La justice sociale, c'est de faire en sorte que le travail paye. « Avec le Président de la République, nous avons reçu cinq sur cinq le message d'exaspération fiscale que les Français nous ont adressé. Ceux-ci ne veulent plus des mots ; ils veulent des actes. Nous avons donc décidé une baisse d'impôts historique : au total, les impôts des ménages baisseront durant ce quinquennat de 27 milliards d'euros. Je vous confirme que la taxe d'habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée pour l'ensemble des Français. » Quand Les 80 % de Français les plus modestes bénéficieront dès ce mois de septembre de la suppression du deuxième tiers de la taxe d'habitation et leur taxe sera intégralement supprimée en 2020. Pour les 20 % de Français restants, la suppression se déploiera sur trois années. « Nous réformerons le financement des collectivités territoriales, en garantissant leur autonomie financière et le dynamisme de leurs ressources. Jacqueline Gourault et Gérald Darmanin reprendront les concertations avec les associations d'élus dès la semaine prochaine. Comme je m'y suis engagé, l'ensemble des mesures devra figurer dans le projet de loi de finances afin de garantir la visibilité aux maires. Nous avons choisi de concentrer l'intégralité de la baisse de l'impôt sur le revenu annoncée par le Président de la République sur les classes moyennes qui travaillent. Le taux d'imposition de la première tranche de l'impôt sur le revenu, qui regroupe 12 millions de foyers, sera abaissé de 3 points. Cela représente un gain moyen par foyer de 350 euros, soit, à ce niveau, un tiers de l'impôt en moyenne. C'est massif, c'est clair, c'est net. Les 5 millions de foyers de la tranche suivante bénéficieront d'un gain moyen de 180 euros. Ces baisses seront votées dans le projet de loi de finances pour 2020. Soyons clairs : baisser les impôts de 5 milliards d'euros, en une fois, nous obligera à faire des choix pour contenir nos dépenses publiques. Certains opposent parfois ceux qui seraient attachés aux équilibres budgétaires à ceux qui feraient vraiment de la politique. Je crois profondément le contraire. La responsabilité politique, c'est de mettre en oeuvre des principes et, en même temps, de respecter le réel. « C'est le choix d'une grande nation, qui veut maîtriser son destin. C'est la marque des Premiers ministres qui m'inspirent. Je pense à Pierre Mendès France et Georges Pompidou, à Michel Rocard et Alain Juppé. » Quelle Le réel, c'est souvent nos sous. Ceux des Français. Ceux que nous prenons pour financer nos politiques publiques ou la redistribution. Ceux de nos enfants, car les dettes que nous créons, ce sont nos enfants qui les rembourseront. Le Président a, dans cette perspective, annoncé la révision de certaines niches fiscales et sociales. Nous nous concentrerons sur les niches anti-écologiques, les niches concentrées sur les très grandes entreprises, ... Total ! ... ou sur les niches qui en fait réduisent les droits sociaux des salariés, comme la déduction forfaitaire spécifique. Dans chacun de ces secteurs, la concertation a montré que le changement était possible, mais qu'il devait être progressif. Nous avons appris de la taxe carbone, et nous ferons donc ces réformes en laissant aux entreprises le temps de s'adapter. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin indiqueront au début du mois de juillet les choix du Gouvernement. La justice, c'est de mieux associer les salariés aux résultats de l'entreprise, de renouer avec l'idée gaullienne de participation. La prime exceptionnelle de fin d'année qu'avait annoncée le Président de la République sera reconduite pour un an en 2020, ... Très bien ! ... avec le même régime défiscalisé dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire. Pour que cet élan soit pérenne, les entreprises devront, pour verser la prime exceptionnelle, mettre en place un dispositif d'intéressement au profit de leurs salariés avant le 30 juin 2020. Nous les y aiderons, en simplifiant la mise en place des accords d'intéressement dans les PME, en les autorisant à tester ces accords sur un an au lieu de trois, en mettant à la disposition des PME des accords-types opposables à l'administration. « La justice sociale, c'est de renouer avec la méritocratie républicaine, avec l'égalité des chances. Trop souvent, notre modèle social repose sur des politiques de compensation qui lissent les inégalités sans chercher à les réduire à la base. La France est un des pays les plus redistributifs au monde et pourtant l'un des pays où le déterminisme social est le plus élevé. Les études PISA montrent par exemple que l'influence du milieu social sur les performances scolaires

Nous irons encore plus loin dans le traitement des difficultés à la racine, en rendant l'école obligatoire dès trois ans, en étendant l'effort de réduction du nombre d'élèves à la grande section de maternelle dans les zones les moins favorisées

les contours d'un nouveau service public d'accueil des enfants handicapés à l'école. Nous voulons en finir avec des systèmes qui bricolent des solutions pour les enfants en situation de handicap, qui trop souvent font leur rentrée après les autres enfants. Nous poursuivrons la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur. Avec la réforme de Parcoursup, que Frédérique Vidal a conduite, les jeunes Français choisissent désormais leur voie par vocation, non plus par défaut », avec la fin de cette absurdité du tirage au sort. Cette réforme qu'on disait impossible, elle est faite, elle marche et elle est juste. » Oh ! « On compte déjà 30 % de plus de boursiers dans les classes préparatoires parisiennes, et les IUT ont admis 19 % de bacheliers technologiques de plus. » Voilà la meilleure réponse aux critiques faites l'année dernière Renforcer notre modèle social, c'est en combler les failles, c'est l'adapter aux situations individuelles, c'est inventer de nouvelles solidarités.

Logement, travail, fins de mois, garde d'enfants : tout est plus difficile quand on est seul. C'est pourquoi, dans le plan Pauvreté, nous avons prévu l'ouverture de 30 000 places en crèches et la formation de 600 000 professionnels. Un service unique d'information des familles sera créé en 2020 pour connaître en temps réel les places de crèches et d'assistantes maternelles disponibles. « Enfin, dès juin 2020, le Gouvernement mettra en place un nouveau système pour protéger les personnes seules contre le risque d'impayés des pensions alimentaires. Sur décision d'un juge, ou sur demande en cas d'incidents de paiement, les pensions seront automatiquement prélevées par la Caisse d'allocations familiales pour être versées à leurs bénéficiaires,

de la tension, de la précarité et laisser les familles seules face à l'incertitude sur le versement des pensions. « Je pense à notre système de soins.

de la lutte contre les discriminations et contre les violences. « Je pense aux millions d'aidants qui arrêtent de travailler ou qui réduisent leur activité pour s'occuper d'un proche. Nous demanderons aux partenaires sociaux de se saisir de cette question, et nous examinerons comment prendre en compte ces situations dans le calcul des retraites. Je pense à tous ceux qui sont perdus face à la complexité de notre système d'aides sociales et pour lesquels nous sommes en train de préparer le futur revenu universel d'activité. La concertation a commencé

C'est l'un de nos grands défis de société. Certains parlent d'une révolution de la longévité ... Nous avons trop tardé pour nous y confronter, parce que les budgets en jeu sont gigantesques, mais aussi peut-être par une forme de déni. Nous le voyons tous avec nos parents ou nos grands-parents : malgré le dévouement des soignants, des familles et des aidants, nous sommes mal préparés. C'est notre regard qui doit changer, celui que nous portons sur la place des personnes âgées dans notre société, le rôle qu'elles peuvent y jouer. Nous devons aussi entendre leur volonté de vieillir à domicile ; entendre les familles qui supportent une charge financière importante et qui souvent sont prises en tenaille entre leurs obligations d'enfants et celles de parents, voire de grands-parents entendre les personnels, dont le métier doit être revalorisé. « La ministre des solidarités et de la santé présentera à la fin de l'année un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous enclencherons une première étape, avec des mesures favorisant le maintien à domicile et des investissements dans les Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Cela fait dix ans qu'on promet cette grande réforme de dignité et de fraternité. Nous la conduirons, et ce sera un autre grand marqueur social de ce quinquennat- peut-être un des plus importants. « L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système universel de retraites. Nous avons aujourd'hui quarante-deux régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite : la France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est supérieur à celui de la population. Cependant, notre système n'est ni simple ni juste. Il pénalise les carrières courtes ou hachées. Ce constat est connu. S'y ajoutent des inquiétudes légitimes concernant son avenir. « Le haut-commissaire Le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye a mené un intense travail de concertation. Il présentera en juillet ses recommandations en faveur d'un système universel permettant à la fois de renforcer l'équité entre générations, la protection des plus fragiles et la confiance des Français. « Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple

entre les pensions des plus modestes et celles des plus aisés, entre les pensions des hommes et celles des femmes. Il garantira enfin, comme le Président l'a demandé, que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85 % du SMIC. « Nous Nous savons tous que ces principes sont justes, mais qu'ils nécessitent des évolutions profondes. S'agissant des fonctionnaires, par exemple, dont les retraites sont calculées actuellement sur les six derniers mois hors primes, le nouveau mode de calcul, sur l'ensemble de la carrière et sur l'ensemble de la rémunération, devra nous conduire à revaloriser les profils de carrière de certaines professions ; je pense en particulier aux enseignants. Les mêmes règles pour tous, c'est vrai, cela signifie aussi la fin des régimes spéciaux. Cela se fera très progressivement, sans modifier les conditions de départ des personnes qui ont déjà des projets pour leur retraite et en conservant l'intégralité des droits acquis. Ce qui compte, c'est la cible vers laquelle nos régimes vont converger ; pour aller vers cette cible, il faut du temps et de la souplesse. Nous nous en donnerons pour réussir cette transformation. Enfin, le Président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. C'est la clé de la réussite du pays. Je vois bien que cela inquiète. Mais, la réalité, c'est qu'il s'agit aussi d'une question de justice. Continuer à partir à la retraite deux ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens, c'est demander à nos enfants de financer cet écart. Et les Français sont lucides déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal, parce que nos compatriotes ont compris que, grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension, et ils ont raison. « Nous maintiendrons la possibilité d'un départ à soixante-deux ans, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix, en liberté et en responsabilité. La condition pour que ce choix existe, c'est que le chômage recule, et c'est la raison pour laquelle nous lancerons un grand plan pour l'emploi des seniors. L'acte II, c'est aussi répondre à un certain nombre de peurs ; des peurs qui se sont exprimées durant le grand débat, qui s'expriment depuis des années dans le débat public. Toutes reposent sur un sentiment de " perte de contrôle " : perte de contrôle sur les évolutions du monde, sur le progrès technologique, sur des menaces réelles ou ressenties, sur la violence. « Il existe plusieurs manières d'appréhender ces inquiétudes ou ces peurs. On peut les attiser pour en tirer profit. On peut les nier, pour éviter de se poser des questions difficiles. Ou, alors, on peut les affronter, en montrant à nos concitoyens que, sur tous les sujets, la République a les moyens de garder le contrôle. « Garder le contrôle, c'est d'abord garantir l'ordre public pour tous et sur tout le territoire. Une de nos premières décisions a été de lancer un vaste plan de recrutement et d'équipements des forces de l'ordre et d'y accorder les moyens. Il y avait urgence, et on partait de loin. Une autre décision a été de concentrer les forces dans les quartiers de reconquête républicaine où la délinquance, les incivilités avaient grimpé en flèche.

notre priorité sera de combattre le trafic de stupéfiants, qui gangrène des pans entiers de notre territoire. Cela implique de harceler les points de vente, de neutraliser les échelons de distribution, de faire tomber les têtes de réseaux. Nous procéderons aux changements d'organisation nécessaires pour parvenir à ces résultats opérationnels. « J'ai également demandé à Christophe Castaner un plan pour lutter contre la violence gratuite. Les Français n'en peuvent plus des coups de couteau donnés pour un mauvais regard ou des batailles rangées entre bandes rivales. Nous ne devons plus rien laisser passer. « Pour réussir, nous devrons finaliser les réformes que nos forces de l'ordre attendent depuis longtemps ... Avoir plus de policiers ! ... sur le temps de travail, sur les heures supplémentaires, sur la fidélisation dans les postes et les territoires. Pour traduire ces orientations, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État engageront, dès cet été, la rédaction d'un Livre blanc sur la sécurité intérieure ainsi que d'une future loi de programmation. Garder le contrôle, c'est maintenir une vigilance de tous les instants contre la menace terroriste, c'est continuer de fermer les lieux de culte radicalisés, c'est poursuivre l'expulsion systématique des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui figurent au FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste- nous en avons expulsé plus de 300 au cours des dix-huit derniers mois c'est poursuivre les efforts de recrutement dans le renseignement : il y en aura 1 900 d'ici la fin du quinquennat. « Garder le contrôle, c'est affirmer notre singularité et notre indépendance dans le monde ; un monde qui est dangereux, où la France, inlassablement, cherche à porter la voix de la paix et de la stabilité en continuant de promouvoir le multilatéralisme contre la loi du plus fort ; en investissant dans l'aide au développement. » Très bien ! « Au-delà des moyens en hausse que nous y consacrons, que nous y consacrons, pour aller jusqu'à 0,55 % du produit intérieur brut, c'est l'ensemble de notre dispositif qui doit être revu. Une mission est en cours, et je sais que les commissions parlementaires ont fait de nombreuses propositions. Le Président de la République tiendra un conseil du développement en juillet et, à l'issue des rencontres du G7 cet été, Jean-Yves Le Drian préparera un projet de loi qui sera déposé au Parlement à l'automne et discuté en 2020. La France doit également rester capable de se battre contre ses ennemis : en Syrie, où la fin du califat territorial est une victoire, mais ne marque pas la fin de la menace au Mali, aux côtés de nos alliés. Je sais que vous vous associerez tous à l'hommage que je veux rendre à celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre. Mes pensées Mes pensées vont à leurs familles, et plus particulièrement à celles qui ont été endeuillées cette année. « Conformément aux engagements du Président de la République, mon gouvernement a voulu donner les moyens à nos armées de nous défendre. Le 13 juillet dernier, le Président a promulgué la loi de programmation militaire pour porter notre effort de défense à 2 % du produit intérieur brut. C'est un effort massif. Mais il s'agit là aussi d'être constant et cohérent. Combattre les peurs du pays, montrer que nous gardons le contrôle, c'est avoir le courage d'affronter sans fausse pudeur certaines réalités, notamment concernant la pression migratoire. Cette réalité, c'est un nombre de demandeurs d'asile qui a baissé de 10 % en Europe l'année dernière, mais qui continue d'augmenter en France de 22 %. » Pourquoi ? « Si nous voulons bien accueillir et bien intégrer ceux qui rejoignent notre pays, nous devons maîtriser ces flux migratoires. « Ce combat est évidemment d'abord européen. Le Président de la République l'a annoncé la France portera dans les prochains mois, avec de nombreux partenaires européens, un projet de refondation complète de Schengen. « Nous devrons également prendre nos responsabilités au niveau national. Le droit d'asile est un trésor. Nous y consacrons des moyens en forte hausse. C'est le prix de la fidélité à nos valeurs, mais c'est aussi pour cette raison que nous devons lutter avec fermeté contre des abus. Nous continuerons évidemment à offrir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et de protection sociale conformes à nos principes. Mais nous devons nous assurer que les demandeurs d'asile choisissent la France pour son histoire, pour ses valeurs, pour sa langue, et non parce que notre système serait plus favorable que celui d'autres pays européens. » Mais c'est c'est que ces sujets devraient faire l'objet d'une harmonisation complète dans l'Union européenne. « Ces questions sont difficiles. Elles soulèvent les passions. Elles touchent aux fondements de notre souveraineté et de nos principes. Il est donc nécessaire d'en débattre de manière régulière et au grand jour avec le Parlement. C'est pourquoi, comme l'a annoncé le Président de la République, le Gouvernement organisera chaque année un débat au Parlement sur les orientations de la politique d'immigration et d'asile. Le premier aura lieu au mois de septembre prochain. Combattre les peurs, c'est lutter contre l'islamisme et faire vivre la laïcité. « Le Gouvernement accompagnera les musulmans dans la construction d'un islam où les croyants français exercent les responsabilités. Nous ne le ferons pas à leur place, mais nous leur donnerons les moyens : d'abord, de combattre l'islamisme et les discours de haine sur les réseaux sociaux- je salue la proposition de loi de Laetitia Avia, qui nous donnera les outils nécessaires ensuite, de réformer l'organisation du culte musulman. Des assises territoriales de l'islam de France ont eu lieu l'été dernier. Un large consensus s'est dégagé en faveur d'une structuration départementale. Il est important que des suites soient données à ces attentes. l'islam de France doit recruter et former des imams en France, qui parlent le français, et mettre fin de manière progressive au système où beaucoup d'imams ou psalmodieurs sont choisis et rémunérés par des États étrangers. S'il faut des dispositions législatives pour garantir le respect de l'ordre public et renforcer la transparence du financement des cultes, en particulier quand ce financement est étranger, le Gouvernement vous les proposera, sans remettre en cause la loi de 1905 ni le libre exercice des cultes. « Combattre les peurs, c'est " remettre de la conscience dans la science ", pour paraphraser une formule célèbre. C'est déterminer ce qui est permis et ce qui ne l'est pas dans des domaines où tout devient techniquement possible. « Les États généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le Gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du Président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions, comme l'accès aux origines, le régime de filiation en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, plusieurs options étaient possibles, et le Gouvernement a retenu celles qui lui semblaient les plus à même de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en conseil des ministres fin juillet et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire. J'ai la chance d'avoir dans mon gouvernement trois ministres d'exception ... Et les autres alors ? ... une médecin, Agnès Buzyn, une juriste, Nicole Belloubet, et une scientifique, Frédérique Vidal. Les débats que vous avez eus avec elle, que j'ai eus avec elles, ont été de grande qualité. Je suis persuadé que nous pouvons atteindre une forme de consensus sur ces dossiers. C'est mon ambition en tout cas. « Combattre les peurs, enfin, c'est regarder l'avenir avec confiance, investir dans l'intelligence, renouer avec l'esprit de conquête. « L'État, qui devrait raisonner en stratège pour le long terme, est trop souvent englué dans le court terme, dans la gestion politique à six mois, alors que des entreprises ou des collectivités territoriales déploient des plans d'action à dix ans, investissent, motivent leurs collaborateurs, cherchent, découvrent. Il faut, comme le Président nous y a invités, tracer une perspective collective de long terme pour notre pays, donner de la visibilité à chacun sur les objectifs de la Nation à l'horizon 2025 bâtir un pacte productif ; rattraper notre retard en robotique, comme nous sommes en train de rattraper notre retard en numérique ; devenir le principal hub de l'intelligence artificielle en Europe ; devenir en tout point la Nation la plus attractive, pour le tourisme, la santé, l'industrie Offrons à la jeunesse des raisons de s'engager, pour l'environnement, pour le développement, dans les territoires isolés, le service national universel, que nous commençons à déployer cette année. « Définissons une nouvelle ambition pour la recherche et l'enseignement supérieur. Je vous saisirai d'un projet de loi de programmation et de réforme au printemps 2020. « Combattons les peurs, le repli, et défendons ce que le Président de la République a appelé " l'art d'être Français ", c'est-à-dire aussi l'art tout court, la culture. Nous poursuivrons le déploiement du pass culture. Nous réaffirmerons, dans le cadre du projet de loi audiovisuel, qui sera discuté au Parlement au tout début 2020, le rôle de l'audiovisuel public dans la diffusion de la culture. Nous défendrons le patrimoine national ; un patrimoine avec lequel, on l'a vu lors de la catastrophe de la cathédrale de Notre-Dame, les Français entretiennent un rapport fort et intime. L'acte II se joue enfin dans la réforme de l'État, non pas au sens bureaucratique qu'on lui donne souvent, mais au sens qu'on lui donnait en 1935, en 1958, quand, déjà, la République cherchait à renouer avec le peuple. « J'ai déjà évoqué, devant vous, le " mur de défiance " qui s'est élevé, au fil des années, entre les Français et ceux qui les représentent ou qui les administrent. J'ai aussi fait le constat avec vous du besoin de proximité et de participation qui s'est exprimé lors du grand débat. Nous ne répondrons pas à ces attentes avec de simples aménagements. C'est l'ensemble de l'action publique- " du sol au plafond ", si vous me permettez l'expression -qu'il faut désormais transformer. « Il y a un an, nous avions présenté un projet de loi constitutionnelle et deux projets de loi complémentaires, organique et ordinaire. Vous comprendrez que je reprenne mon souffle sur ce sujet ... « Les circonstances n'ont pas permis leur examen,

nous ont confortés dans notre conviction que ces textes étaient utiles, et le grand débat nous a permis de les enrichir.

reprennent le coeur des engagements du Président de la République, y compris l'inscription de la lutte contre le changement climatique à l'article 1 de notre Constitution. Ils sont recentrés sur trois priorités les territoires, avec l'autorisation de la différentiation, l'assouplissement du cadre relatif à la Corse ainsi qu'aux outre-mer la participation citoyenne, avec un nouveau titre dans la Constitution, la transformation du Conseil économique, social et environnemental en conseil de la participation citoyenne, la possibilité de former des conventions de citoyens tirés au sort, la facilitation du recours au référendum d'initiative partagée et l'extension du champ de l'article 11 ; la justice, avec l'indépendance du parquet et la suppression de la Cour de justice de la République. En parallèle, des gestes ont été faits pour parvenir à un consensus avec le Sénat. » Lesquels ? « Les dispositions relatives au fonctionnement des assemblées ont été retirées. Nous avons considéré qu'il appartenait aux assemblées elles-mêmes de décider de leurs réformes. » C'est sûr ! Très bien ! « Les dispositions relatives au cumul des mandats dans le temps ont été assouplies pour en exclure les maires de communes de petite taille et prévoir une entrée en vigueur progressive. Le Président de la République la République a accepté de revoir sa proposition de baisse d'un tiers du nombre de parlementaires pour viser une réduction d'un quart, qui permet une juste représentation territoriale et l'introduction d'une dose significative de proportionnelle. » Quel silence ! « La réalité, aujourd'hui, c'est que nous sommes proches d'un accord sur le projet de loi constitutionnelle, mais que ce n'est pas encore le cas sur le projet de loi organique, ... Non plus ! ... et en particulier sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Et le Sénat a été très clair sur le fait qu'il n'y aurait d'accord sur rien s'il n'y avait pas accord sur tout.

et la manifestation de volonté du Sénat, qui, peut-être, ne viendra qu'après le renouvellement de la Haute Chambre en 2020. Nous pouvons aussi voter seulement la proportionnelle à l'Assemblée nationale,sans changer le nombre de députés. Et le Président de la République ala faculté d'interroger directement les Français sur la réduction du nombre de parlementaires. Ma conviction est que nous ne devons pas résister au désir de changement exprimé par les Français. » Les gens

j'ai signé deux instructions qui remodèlent nos administrations, à Paris et sur le terrain. Dès janvier prochain, 95 % des décisions individuelles seront prises sur le terrain.

Les services locaux seront renforcés, réorganisés pour plus de cohérence, les administrations centrales allégées et rendues plus agiles. « Dans le même temps, nous achèverons d'ici l'été l'examen de la loi de transformation de la fonction publique, et nous donnons plus de pouvoir aux managers. La mission Thiriez démarre ses travaux sur la haute fonction publique, pour rénover profondément son recrutement, sa formation et la gestion des carrières. C'est un dossier déterminant pour l'État, parce que pouvoir bénéficier des meilleurs éléments, et des plus dévoués, a toujours été essentiel. Je m'en occuperai personnellement. Le service public, c'est une promesse républicaine, en particulier pour les territoires isolés, la ruralité, les quartiers, l'outre-mer. Des personnes, un accueil, un conseil

Depuis plusieurs années, les maisons de services au public ont tenté d'apporter une première réponse. Certaines le font déjà remarquablement. Je l'ai vu à Montmoreau, en Charente. Mais reconnaissons ensemble que les maisons de service public sont très variées et proposent des niveaux de service très différents. Nous devons changer d'échelle et de logique partir des besoins de nos concitoyens, dépasser les frontières des administrations, oublier que nous sommes l'État, le département, la Caisse primaire d'assurance maladie ou la Caisse d'allocations familiales. Cela veut dire des choses simples, comme des horaires d'ouverture élargis, des agents polyvalents, capables d'offrir immédiatement des réponses, d'accompagner vers la bonne porte d'entrée.

J'aurai également le plaisir de signer avant le 14 juillet les contrats de convergence et de transformation avec les collectivités ultramarines des contrats qui mettent en oeuvre nos objectifs de développement économique et social dans ces territoires et qui s'inscrivent résolument dans la transition écologique. Je veux redire, comme je l'avais fait lors de ma première déclaration de politique générale, à nos compatriotes ultramarins notre volonté de faire appliquer en toutes circonstances ce que j'ai appelé un " réflexe outre-mer ". Nous tiendrons nos engagements. « Transformer Transformer l'action publique, enfin, c'est répondre à l'aspiration fortement exprimée dans le grand débat pour plus de simplicité et plus de proximité. Je suis favorable, pour ma part, à un nouvel acte de décentralisation, mais je sais que cela prend du temps et que les positions des territoires sont moins unies que nous ne le voudrions tous. C'est C'est bien normal, d'ailleurs, car notre système est devenu compliqué. « Ma conviction, c'est qu'il faut d'abord conforter les maires, qui sont plébiscités par nos concitoyens, pour répondre au sentiment de fracture territoriale. « Je vous propose donc de procéder en deux temps. D'abord, en prenant des mesures pour favoriser l'engagement des maires. Elles seront rassemblées dans un projet de loi que le Gouvernement présentera dès le mois de juillet et que je proposerai au Sénat d'examiner dès la rentrée. normal, c'est la Constitution ! « Ensuite, nous devrons nous accorder avec les élus et leurs représentants sur la meilleure méthode pour clarifier le fameux " millefeuille territorial Il faut aller vers des compétences clarifiées, une responsabilité accrue, des financements clairs, comme le Président de la République nous y a invités. » Depuis le temps qu'on entend ça ! « J'irai demain solliciter l'approbation de la politique du Gouvernement au Sénat. Mes prédécesseurs l'ont peu fait, et encore, seulement lorsque le Sénat était clairement dans la majorité.

sans penser revenir avec une majorité. Mais ce sera l'occasion pour le Gouvernement de détailler ce chapitre territorial de l'acte II, et le vote permettra

j'ai appelé au dépassement pour relever les défis, mais je reconnais que le Gouvernement aussi doit dépasser ses habitudes, ses inclinations, pour changer de méthode. Le sentiment d'urgence nous a parfois conduits à prendre des décisions rapides, pas assez concertées. » C'est vrai ! « C'est toujours une erreur et, au final, cela fait perdre du temps. Dans ma vie de maire, j'ai pu constater qu'écouter c'est toujours mieux pour se faire entendre. « En cette troisième année aux responsabilités, nous voulons faire évoluer notre manière de gouverner. Nous sommes et nous demeurerons des réformateurs, mais nous devons davantage associer les Français à la fabrique de nos décisions. Les transformations que nous avons engagées,

Je pense notamment aux retraités et aux Français des territoires isolés. C'est à nous de les convaincre que nous les faisons pour eux, ... Ça va être dur ! ... à nous de changer de méthode pour les faire avec eux. C'est le sens de la mobilisation nationale qui réunit sur les territoires élus, partenaires sociaux, associations, services de l'État, pour identifier ce qu'on doit changer au service de l'emploi et de la transition écologique. C'est le sens aussi du développement d'une forme de démocratie directe »- et participative -, « parce que le grand débat n'est pas une parenthèse, mais un besoin de fond de nos démocraties. Le sens enfin de cette attention que nous devons apporter à ce " fameux dernier mètre " qui sépare parfois une décision prise dans un lointain bureau ministériel des Français, qui, seuls, comptent. Changer de méthode, c'est aussi changer de ton. La détermination, la conviction, la passion que nous mettons à défendre nos idées ne devraient jamais nous conduire à l'arrogance, à l'agressivité, à la caricature.Regardons avec lucidité notre scène politique et nos débats médiatiques. Ils ne sont pas toujours à la hauteur des enjeux. Je ne donne aucune leçon, ... Vous ne faites que ça ! ... et je ne m'exonère d'aucune responsabilité dans ce domaine, mais nous avons à traiter de belles questions, qui méritent mieux que des raccourcis, des outrances ou des postures. Ces belles questions méritent, elles aussi, que nous dépassions nos vieilles habitudes ; que nous nous écartions de ces partitions vieillies qui nous font jouer, mal le plus souvent, les mêmes rengaines fatiguées. » On n'est pas à la maternelle ! La France, qui est souvent belle dans la tradition et la permanence, n'est jamais aussi grande que dans l'effort et le dépassement. Dans le pays des Lumières, ce n'est jamais l'argument d'autorité qui doit prévaloir ; dans le pays des Lumières, on doute et on se respecte. Je ne me résigne pas au rétrécissement du débat public, et je souhaite que nous portions ensemble l'espoir d'un ressaisissement, sans gommer nos différences. Il est un joli mot, qui vient de la rude et grave républicaine romaine, mais qui semble parfois faire défaut dans nos démocraties, c'est celui de " civilité " une civilité qui va au-delà de la politesse de façade et qui concerne, au fond, le respect que l'on doit à tout membre d'une même communauté. Si vous le voulez bien, c'est, après le dépassement, le second terme que j'aimerais placer au coeur de notre projet, pour marquer le respect, la considération que chacun a le droit le plus fondamental de revendiquer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, notre feuille de route est claire pour l'année qui vient, mais notre vision pour le pays va bien au-delà d'une année de travail, aussi intense soit-elle. Nous souhaitons réconcilier la France avec elle-même. Notre pays, qui a tout et que le monde envie, a perdu confiance. En tout cas, des millions de ses citoyens ont perdu confiance en lui. Cette confiance, nous voulons la rebâtir, en renouant avec l'idée de rassemblement, car notre pays a besoin d'unité et de respect, en renouant avec l'idée de puissance, gage de notre grandeur et de nos modes de vie, modes de vie, en remettant l'humain au coeur de nos préoccupations. « Une France fidèle à elle-même, puissance industrielle, militaire et culturelle, une France travailleuse, solidaire et écologique, qui puise dans ce qu'elle produit la ressource de la justice sociale et qui ne vit pas au crédit de ses enfants, ni de leur environnement. Je me tiens devant vous pour tenir les engagements du Président de la République et mettre fidèlement en oeuvre l'intégralité de ce que je viens de vous annoncer. Et j'ai l'honneur d'engager

de dire, chers collègues, monsieur le ministre,

une injure à tous ces hussards de la République honorés de se dévouer gratuitement pour nos communes, à en croire les croyants, non pratiquants d'ailleurs, de cette morale très exigeante. Nous allons voir si les temps sont venus de mettre fin à cette hypocrisie séculaire : reconnaître que la commune est le terreau de la République et de la démocratie françaises, le premier garant de la cohésion sociale, le premier pourvoyeur de services publics de proximité, le premier investisseur public et, directement ou indirectement, le deuxième employeur public ; et, en même temps,

Un statut, en effet, fixe l'ensemble des garanties et des obligations qui, s'attachant à une personne, à un groupe, à un territoire, les distingue des autres, facilitant ainsi l'accession du plus grand nombre aux fonctions électives, sans préjudice professionnel ou financier, et permettant la représentation de la population dans toute sa diversité. Instituer un tel statut serait prendre au sérieux notre Constitution, laquelle donne un fondement politique aux institutions locales. Selon les termes de celle-ci, « l'organisation » de la France est « décentralisée »- c'est l'article 1 - ; « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon » et elles « s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences »- c'est l'article 72. Les communes sont donc loin d'être des institutions destinées à donner un vernis démocratique à une administration d'État déconcentrée ou, encore moins, à offrir un passe-temps à des notables rentiers. Prendre au sérieux l'idée de décentralisation, reconnaître symboliquement l'importance de la mission de ceux qui administrent et donnent vie à la commune, ce que fait d'ailleurs la loi fondatrice de la nouvelle décentralisation du 2 mars 1982, qui prévoyait déjà une loi instituant un statut de l'élu local. Celle-ci sera semi-enterrée sous les couches de projets et propositions destinés à « améliorer » ou « faciliter » telle ou telle « condition d'exercice des mandats locaux

que « les fonctions de maire, d'adjoint et de membre du corps municipal sont essentiellement gratuites ». Par ailleurs, aux termes de cette loi, « aucun électeur ne pourra déposer son vote qu'après avoir prêté entre les mains du président serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constitutionnelle et aux lois du royaume ». Étrange hommage de la République à la Monarchie de Juillet ! Accessoirement, supprimer l'article L. 2123-17 du code général des collectivités permettrait de sortir du dilemme qui fait actuellement des indemnités de fonction soit le salaire d'une fonction publique croupion- c'est le cas du rapport Mauroy de 2000 -, soit une forme de dédommagement soumis à impôt et à cotisations sociales, ce qui n'est pas banal pour un dédommagement. Un dédommagement d'on ne sait quoi- perte de revenu même si on est retraité, frais divers ... -cohabitant avec la compensation de frais annexes, comme les frais de représentation Tout cela resterait une entorse à la logique si, de glissement en glissement, « l'indemnité » n'était pas devenue pour Bercy un salaire comme les autres, imposable selon les modalités communes, et pour les percepteurs sociaux un revenu à taxer comme les autres. Ainsi l'article 10 de la loi de finances pour 2017, sans crier gare, supprimait-il la possibilité de déclaration fiscale séparée des indemnités électives et des autres revenus, entraînant de fait une majoration importante de l'impôt pour nombre d'élus : « Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux en application du code général des collectivités territoriales sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles

outre la valeur symbolique de la reconnaissance de la fonction communale, instituer un statut de l'élu municipal est le seul moyen d'endiguer la dérive qui fait de l'élu territorial, et particulièrement communal, dans l'exercice de ses fonctions, fonctions, exercées- je le rappelle -au nom de la collectivité et dans l'intérêt général, un simple citoyen ou un professionnel. En effet, si la longue liste des responsabilités des élus n'a rien à voir avec celle du citoyen lambda ou même d'un chef d'entreprise, d'un médecin ou d'un avocat, il en va différemment de sa responsabilité pénale. Au mieux, elle est la même ; souvent, elle est plus lourde, au motif que l'intéressé est « investi d'un mandat électif public », d'un pouvoir général de police ou « dépositaire de l'autorité publique ». Le meilleur résumé de la situation nous est donné par Camille et Jean de Maillard Maillard : aujourd'hui, « on n'est plus citoyen que pour s'abstenir d'agir, à moins de vouloir assumer une responsabilité dont on devient l'infamant débiteur Tant qu'on refusera d'articuler principe d'égalité devant la loi et réalité de l'inégalité devant les charges, responsabilités et obligations, ce qui devrait être au coeur d'un authentique statut de l'élu territorial, on en restera là Tant qu'il y aura évidemment des amateurs au rôle « d'infamant débiteur ». Trois urgences : préciser les notions de « prise illégale d'intérêts » et de « délit de favoritisme », ce que le Sénat a déjà fait à l'unanimité à trois mais qui a disparu dans le trou noir de la navette ; préciser l'article 122-4 du code pénal en donnant force de loi à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 octobre 2012 relaxant le maire de Cousolre, dans le Nord, précédemment condamné pour avoir donné une gifle à un adolescent provocateur. Mais l'institution d'un statut de l'élu communal ne saurait se limiter à une reconnaissance des responsabilités particulières particulières des administrateurs communaux élus et à l'amélioration des conditions d'exercice de leur mandat. Elle doit aussi préciser les droits des conseillers municipaux, tout particulièrement ceux de l'opposition, trop souvent tributaires de la bonne ou mauvaise volonté du maire et de sa majorité. Pour que la commune soit réellement la « cellule de base » de la démocratie, il faut que ce soit un lieu réel de débat informé sur un pied d'égalité. Avant de succomber aux charmes imaginaires de la démocratie « post-représentative l'urgence est pour moi de revivifier la démocratie représentative, en donnant toute sa place à un débat démocratique trop souvent réduit à l'exposé de discours parallèles- pour ne pas dire à un dialogue de sourds. La démocratie, avant d'être le pouvoir des majorités, c'est d'abord le débat démocratique à égalité d'information. Tel est l'esprit de cette proposition de loi, qui évidemment aborde aussi l'ensemble des dispositions pratiques susceptibles d'améliorer les conditions d'exercice des mandats municipaux : disponibilité des élus, formation, sécurité matérielle, professionnelle et juridique pour s'en tenir à l'essentiel. À vous de dire, chers collègues, monsieur le ministre,

chers collègues, la proposition de loi dont le Sénat est saisi aujourd'hui vise à améliorer le statut de l'élu communal. Le législateur se doit en effet d'offrir aux élus les garanties nécessaires pour qu'ils puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions, au service de l'intérêt général. Des évolutions récentes rendent cette préoccupation aiguë : les vagues de décentralisation successives ont augmenté considérablement les responsabilités des élus locaux le droit à appliquer devient de plus en plus complexe, tandis que les services de l'État diminuent leur appui aux collectivités territoriales ; la montée en puissance de l'intercommunalité multiplie les instances auxquelles doivent assister les élus communaux les citoyens sont de plus en plus exigeants envers leurs élus qui sont, comme l'aime à dire le président Larcher, « à portée d'engueulade Résultat : l'exercice d'un mandat local demande toujours plus de temps et d'investissement, alors que les conditions d'exercice des mandats n'ont que faiblement progressé. Le monde du travail évolue aussi, ce qui explique qu'il soit de plus en plus difficile de concilier l'exercice d'un mandat avec la vie professionnelle. la progression de la place des femmes dans les assemblées élues et l'évolution des structures familiales expliquent sans doute le besoin de trouver une meilleure conciliation entre l'exercice du mandat et la vie familiale. Les maires et les autres élus municipaux sont le visage de la République au quotidien. Si nous souhaitons qu'ils continuent à s'engager, il est essentiel d'apporter des réponses à leurs attentes. Notre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation et la commission des lois se sont saisies de ce sujet. La délégation a lancé en décembre 2017 un travail d'ampleur, aboutissant à la conclusion que les conditions concrètes d'exercice des mandats locaux devaient être améliorées, sans que soit remise en cause la conception française de la démocratie locale. J'insiste sur ce point, parce que 17 500 des 35 000 maires ont pris la peine de répondre à la concertation à laquelle ils étaient conviés. a publié le 5 juillet 2018 un rapport en six tomes, abordant chacun des secteurs dans lesquels des améliorations s'avèrent nécessaires. Il s'agit, pour mémoire, du régime indemnitaire, du régime social, de la formation, de la reconversion, de la responsabilité pénale et des obligations déontologiques. Elle a formulé 43 recommandations qui constituent une feuille de route pour les semaines et les mois à venir. Par ailleurs, la commission des lois s'est largement saisie du sujet au travers des travaux de la mission de contrôle et de suivi des lois de réforme territoriale. Cette démarche a abouti à la rédaction d'un rapport visant à revitaliser l'échelon communal, qui porte de nombreuses propositions concernant les conditions d'exercice des mandats locaux. invitons-nous le Gouvernement à s'inspirer sans retenue des apports du Sénat sur ce sujet dans le cadre de ses futurs projets de loi relatifs à la décentralisation et aux élus locaux. C'est donc dans ce contexte que nous sommes appelés à examiner la proposition de loi créant un statut de l'élu communal, présentée par notre collègue Pierre-Yves Collombat et les membres du groupe CRCE et déposée sur le bureau du Sénat le 12 février 2019. Ce texte présente des pistes de réflexion intéressantes, sur des sujets consensuels comme la formation des élus, ou encore la transition entre le mandat local et la vie professionnelle. Je souhaite donc avant tout saluer l'initiative de notre collègue, qui apporte sa contribution à l'un des chantiers les plus déterminants pour l'avenir de nos communes : celui des conditions d'exercice des responsabilités et donc de la vigueur de la démocratie locale. D'une manière générale, sans doute le texte gagnerait-il, afin de tendre vers les objectifs qu'il s'est fixés, à s'enrichir d'un certain nombre de modifications. Au travers des auditions que j'ai menées, j'ai pu relever que certaines mesures prévues dans le texte, si elles tendent à répondre à des besoins avérés, demanderaient davantage d'expertise afin d'évaluer leur impact financier sur les communes et leurs groupements, ainsi que sur les entreprises. Nous savons tous la modestie des moyens dont bénéficient les parlementaires dans le cadre de l'initiative législative et l'extrême difficulté de se livrer à une étude d'impact globale des réformes que nous aimerions apporter au droit existant. Mais certaines dispositions, dont je saisis pleinement l'intention, seraient même difficilement soutenables pour les communes sans une revalorisation très importante des dotations de l'État, sur laquelle nous n'avons malheureusement ici- je le regrette ! -aucune prise. Par ailleurs, certaines divergences peuvent être observées entre les intentions exprimées par l'auteur de la proposition de loi dans l'exposé des motifs et les conséquences en droit des dispositions prévues. Certaines mesures pourraient même avoir des effets contre-productifs-nous y reviendrons. Toutefois, en vertu de la sage coutume pratiquée dans notre assemblée, la commission des lois n'a pas établi de texte et a préféré que la discussion en séance porte sur le texte initial de la proposition de loi. Cela permet de respecter l'intégrité du travail mené par l'auteur tout en permettant, dans le cadre de la séance publique, de faire apparaître clairement les points de convergence et de divergence. Dans cette perspective, la commission des lois a déposé plusieurs amendements visant à modifier, préciser ou compléter, parfois dans l'esprit poursuivi par l'auteur, le contenu de la proposition de loi. Ces amendements s'inscrivent dans la voie étroite laissée à l'initiative parlementaire par les règles constitutionnelles de recevabilité financière, c'est-à-dire l'article 40 de la Constitution, et constituent donc une base de discussion pour aboutir à une amélioration concrète des conditions d'exercice

pas opportunes. Il s'agit notamment des dispositions relatives à la création d'un fonds national pour la formation des élus locaux, dont le dispositif de financement apparaît fragile, et à la création d'une majoration indemnitaire pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer à à leur mandat local ; des dispositions manquant de précision, comme les articles 5 et 6 de la proposition de loi, qui concernent les frais de garde des enfants des et diverses dispositions d'ordre fiscal ; des dispositions qui pourraient alourdir les contraintes pesant sur nos communes, notamment les plus petites d'entre elles. D'autres amendements tendent à corriger tendent à corriger certaines anomalies du droit existant : afin de donner aux conseillers communautaires des communautés de communes les mêmes droits que ceux des conseillers communautaires des autres catégories d'EPCI ou de prévoir une délibération des communes nouvelles dans les trois mois suivant leur création sur les orientations et crédits ouverts au titre de la formation des membres du conseil municipal. Enfin, la commission des lois a donné un avis favorable à plusieurs amendements extérieurs qui complètent utilement le texte. Mes chers collègues, améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux constitue une ardente nécessité, d'autant plus impérieuse que les évolutions actuelles rendent les maires toujours plus vulnérables. Je vous propose donc d'engager une discussion sur ce sujet qui, ici- je le crois, et j'en suis même certain -, nous mobilise tous, afin de confirmer l'engagement de notre assemblée en faveur de cette évolution. Cette discussion pourra nous permettre également d'examiner les points de convergence entre nos positions et celles du Gouvernement. et celles du Gouvernement. C'est d'ailleurs l'une des vertus du texte proposé par notre collègue Pierre-Yves Collombat et les membres de son groupe que de nous offrir l'occasion d'interpeller le Gouvernement à travers vous, monsieur le ministre, pour lui rappeler la vigilance de la Haute Assemblée quant aux engagements qu'il a pris, afin qu'ils ne restent pas lettre morte.

je tiens tout d'abord à remercier le sénateur Pierre-Yves Collombat, à qui je manquais visiblement, qui est à l'initiative de ce texte. On voit bien d'ailleurs, monsieur le sénateur, à la lecture de votre proposition de loi, que de nombreuses mesures s'inspirent directement de votre expérience d'élu local, notamment de maire, dans laquelle je me reconnais moi-même pleinement. Le Sénat s'est rapidement emparé de cette question du « statut de l'élu », même si, je l'ai déjà dit, ce terme ne me paraît pas le plus adéquat pour parler du rôle et de la place qu'occupent les élus locaux dans la République. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, sous la présidence du ministre Jean-Marie Bockel, a notamment travaillé, et de manière très approfondie, sur ce sujet, avec la remise d'un rapport complet visant à « faciliter l'exercice des mandats locaux ». Ce sujet est particulièrement d'actualité, puisque, lors de sa conférence de presse du 25 avril dernier, le Président de la République a clairement rappelé la légitimité des élus, et notamment des maires. Il s'est d'ailleurs engagé à conforter leur rôle, en leur donnant un « statut digne de ce nom ». Ces annonces font, évidemment, suite aux nombreux échanges que le Président de la République a eus avec les maires dans le cadre du grand débat national : les 96 heures de débat en présence de plus de 5 000 élus locaux ont permis, de toute évidence, d'aborder un périmètre encore plus large de sujets. Pendant ces échanges, nous avons entendu un besoin de proximité, de clarté et d'enracinement. Ainsi, après une concertation aussi riche, il est désormais temps de répondre aux nombreuses propositions directement exprimées par les élus, certaines- on peut se le dire -ne datant pas d'hier. C'est tout le sens de la campagne que le Gouvernement va lancer sur l'engagement, afin de redonner à nos concitoyens la possibilité de participer et de s'engager au niveau local, avec une échéance à avoir en tête : les élections municipales de 2020. En effet, je ne vous cache pas mon inquiétude de voir, peut-être pour la première fois dans ce volume, des communes dans lesquelles les listes pour les municipales seront incomplètes, voire pour certaines dans lesquelles aucun candidat au poste de maire ne se déclare. C'est un constat auquel le Gouvernement, tout comme le Parlement, et singulièrement le Sénat, ne peut se résoudre. C'est pourquoi, vous le savez, nous allons porter dans les prochaines semaines un projet de loi autour de cette thématique clé de l'engagement. Cette tribune, monsieur le sénateur Collombat, me permet de vous livrer en avant-première quelques éléments de méthode avant que le Premier ministre n'approfondisse davantage, demain matin avec vous et vendredi avec les maires de France à Albi, le contenu du projet de loi. se structurera, plus particulièrement, autour des trois grandes étapes du parcours d'un élu. Avant l'élection, comment donner envie aux citoyens de franchir le pas et de s'engager dans un mandat local ? local ? Pendant l'exercice du mandat, comment rendre le quotidien de ceux qui se sont engagés plus facile ? En clair, comment ne pas les décourager ? C'est là que les « irritants » de la loi NOTRe doivent trouver des réponses. Après le mandat, dans une société dans laquelle nous avons bien du mal à dire merci à celles et ceux qui se sont engagés, comment les accompagner dans leur reconversion éventuelle ? L'objectif de ce projet de loi est de parvenir à lever les freins à l'engagement qui existent aujourd'hui. Nous souhaitons donc présenter un texte, devant votre assemblée, à la rentrée de septembre, pour une adoption définitive d'ici à la fin d'année, afin qu'il soit effectif pour les élections municipales de 2020. En termes de méthode, je mène depuis plusieurs semaines des concertations étroites avec les associations d'élus, mais aussi naturellement avec les parlementaires. Le Gouvernement souhaite vraiment que ce texte soit réellement coconstruit avec l'Assemblée nationale, mais aussi avec le Sénat. D'ores et déjà, je tiens à remercier les sénateurs avec qui j'ai eu de nombreux échanges, après les propositions de loi de M. Marc et de Mme Gatel, fruits d'un dialogue apaisé avec le président Larcher sur ce projet de loi.

Le Président de la République a également annoncé une nouvelle étape de décentralisation reposant sur trois principes : responsabilité, lisibilité, financement. L'objectif est de redonner davantage de liberté aux élus locaux et de clarifier les compétences et responsabilités de chacun.

En effet, les sujets évoqués dans ce texte s'inscrivent directement dans la lignée des travaux que nous comptons mener. Mais cette proposition de loi, monsieur le sénateur Collombat, arrive, et vous n'y êtes pour rien,

Concernant les mesures proposées dans votre texte, prenons d'abord les propositions qui nous paraissent faire consensus. D'abord, sur la disponibilité des élus, votre proposition d'étendre le congé électif de dix jours aux salariés candidats au conseil municipal des communes de plus de 500 habitants, au lieu de 1 000 aujourd'hui, va de toute évidence dans le bon sens. Plus globalement, je crois qu'il faut poser la question de l'accès des conseils municipaux à des profils qui ne sont aujourd'hui pas suffisamment représentés, comme les salariés du secteur privé. Ensuite, sur la formation des élus, nous sommes globalement en phase avec ce besoin de renforcer la formation, et notamment de l'étendre aux communes de plus de 1 000 habitants, contre 3 500 aujourd'hui. Mais l'enjeu réside aussi dans le financement. Vous proposez la création d'un fonds alimenté par des sommes non dépensées. Cela nous paraît encore un peu prématuré, car créer un fonds dont le montant n'est pas évalué pourrait être contre-productif. il faut surtout réfléchir à son articulation avec les dispositifs existants, sous peine de créer un ensemble peu lisible pour nos collègues élus locaux. Là encore, nous travaillons plutôt à une réforme plus globale de la formation, en essayant de mieux articuler les dispositifs existants, si j'ose dire historiques. Enfin, sur les frais de garde, même même constat : nous sommes d'accord avec la philosophie de votre texte, même si l'article, tel que rédigé, ne convient pas, car il reprend mot pour mot celui qui existe déjà dans le code général des collectivités territoriales. Néanmoins, je peux vous dire que ce sujet aura sa place dans le projet de loi prochainement présenté.

nos collègues élus locaux sont particulièrement attachés, me semble-t-il, à cet esprit ; une indemnité n'est pas un salaire ni un traitement de fonctionnaire.

D'abord, il est important de rappeler que les élus, et peut-être même leurs associations, ne réclament pas systématiquement une hausse des indemnités. C'est une évidence, mais il convient de le rappeler : on ne devient pas élu pour gagner de l'argent.

création de commissions des finances dans les communes de plus de 1 000 habitants, établissement de rapports sur les dépenses de communication du conseil municipal, encadrement des questions orales pour l'opposition. Certaines dispositions, déjà présentes dans le code, sont c'est une conviction personnelle -, plutôt que de tout réglementer et de créer de nouvelles pages pour la prochaine édition du code général des collectivités territoriales, il me semble préférable de faire confiance aux maires et aux élus locaux.

La loi du 31 mars 2015 prévoit d'ores et déjà une possibilité de suspension du contrat de travail pour le salarié du secteur privé, avec une possibilité de réintégration au bout de deux mandats Avant d'aller plus loin, il me paraît important, d'une part, de mener une concertation auprès des organisations professionnelles d'employeurs et, d'autre part, d'avoir une réflexion sur la taille des entreprises ; ce qui est possible pour une grande entreprise l'est peut-être moins pour une TPE, c'est une évidence. En conclusion, je

Je vous propose de continuer ce débat dans le cadre de l'examen des amendements, mais, vous l'aurez compris, à ce stade, le Gouvernement ne peut pas émettre expressément un avis favorable global sur cette proposition de loi. Gageons en tout cas qu'elle fera office d'introduction heureuse aux travaux que nous mènerons ensemble en septembre

Cette proposition de loi de Pierre-Yves Collombat comporte bien des atouts ; le premier est de s'appuyer sur un travail sérieux, le deuxième de prendre en compte l'équipe municipale, le troisième de vouloir réhabiliter d'urgence le rôle du maire, des adjoints, des conseillers et, au travers d'eux, du bloc communal. À quelques mois des municipales, il paraît indispensable que l'avis du Sénat, au travers tant de cette proposition de loi que des travaux de la délégation aux collectivités territoriales, soit pris en compte pour renforcer l'attractivité de l'engagement communal, notamment pour les plus petites communes. Nous le savons tous ici, des élus communaux envisagent sérieusement de jeter l'éponge, tandis que des équipes peinent à se constituer. Sans élu communal- maire, adjoints, équipe volontaire -, il n'y a pas de démocratie de proximité vivante possible. Des habitants qui ne souhaitent plus s'engager, c'est le risque de la fermeture par défaut d'une mairie, de la fusion par défaut avec une autre commune, de l'éloignement par défaut des infrastructures publiques ; mais la démocratie locale, ce n'est pas un défaut, c'est une envie. Une commune sans élus, c'est aussi la disparition d'autres formes d'engagement qui alimentent en permanence la démocratie locale des animations, des réunions publiques, de petits ou de grands débats ; autant de sociabilités qui valent bien mieux qu'un tête-à-tête avec les chaînes d'information en continu ou avec la rancoeur de réseaux sociaux. Je formulerai trois remarques sur le texte même, et un point plus spécifique en conclusion. Première remarque : même si cette proposition de loi désigne l'élu communal en général, c'est bien l'élu des communes de moins de 3 500 habitants et, plus encore, celui des communes de moins de 1 000 habitants qui méritent amplement notre attention. Il n'y a pas de petits élus, mais il y a des élus au service de communes de petite taille.

La décentralisation tient compte de la diversité des territoires ; elle doit aussi tenir compte de la spécificité de ses représentants. C'est pourquoi nous soutenons la revalorisation des indemnités pour les maires et pour les adjoints proposée par ce texte, tout en étant ouverts à la possibilité de la réserver aux élus de communes de plus petite taille. Deuxième remarque : il faut impérativement sécuriser le mandat des élus des petites communes. Sécuriser ne veut pas dire donner un blanc-seing, mais cela signifie prendre en compte l'exercice particulier de certaines missions. Nous sommes ainsi d'accord avec l'objectif de cette proposition consistant à préciser des notions juridiques telles que l'autorité légitime, la prise illégale d'intérêts et le délit de favoritisme. Nous proposons de clarifier la situation des élus en arrêt maladie et exerçant leur mandat, pour éviter qu'ils ne soient obligés, par méconnaissance, de rembourser des sommes importantes. De manière plus globale, nous pensons que les élus, comme leurs administrés, pourraient bénéficier d'un « droit à l'erreur Mes chers collègues, on n'administre pas une commune avec la peur au ventre ; on l'administre avec éthique, avec le souci de bien faire et avec le sens de l'intérêt général. Troisième remarque : nous sommes plus que favorables à ce que le statut d'élu communal soit valorisable et pris en compte dans un parcours de vie. Six ans de mandat mobilisent en effet des compétences professionnelles et relationnelles importantes. Nous proposons plusieurs amendements tendant à préciser que le mandat de maire ou d'adjoint est reconnu par une validation des acquis. Nous soutenons un droit renforcé à la formation professionnelle. Nous souhaitons par ailleurs que ce mandat ne constitue pas un coup d'arrêt dans une carrière antérieure ou un empêchement de progression, dans le public comme le privé. Je soutiens également le fait d'accorder le bénéfice de l'allocation différentielle de fin de mandat aux maires de communes de moins de 1 000 habitants dont le mandat s'arrête. Je demande également des avancées sur le régime d'imposition prévu pour les élus de communes de moins de 1 000 habitants.

Cette reconnaissance est également pour nous un gage supplémentaire de diversification des candidats à la fonction d'élu communal. Plus encore, même si nous connaissons tous des élus communaux disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7- il faut aussi prendre en compte les aspirations de vie, qui sont différentes, des plus jeunes générations. La valorisation des acquis et la formation constituent des réponses intéressantes pour ces vocations.

et plaidé pour une couverture numérique accélérée et des services publics de proximité. C'est surtout la raison pour laquelle notre groupe a proposé la création de l'agence nationale de cohésion des territoires, qui accompagnerait réellement les élus communaux, aiderait à monter des dossiers, éclairerait des procédures tortueuses et rendrait leur gestion quotidienne plus simple et plus juste. Un élu communal sécurisé, pleinement reconnu dans son mandat, n'est pas un élu esseulé ; il travaille main dans la main avec les services de l'État.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons tous été frappés par cette enquête menée par l'Association des maires de France et le Cevipof, selon laquelle 49 % des maires ne souhaitaient pas se représenter aux échéances locales de 2020. Ce nombre atteint même 60 % pour ceux qui réalisent en ce moment même leur premier mandat électif.

avec la vie professionnelle et personnelle, alors que,, la limitation du cumul des mandats appelle davantage de fluidité dans le parcours entre le mandat et la vie professionnelle. Cela

au regard des insuffisances régulièrement soulignées, il est impératif d'améliorer les conditions concrètes d'exercice des mandats locaux, sans que soit remise en cause la conception française de la démocratie locale. Le statut d'élu communal doit permettre de concilier le mandat avec la vie professionnelle et personnelle des élus, de donner à ces derniers les moyens d'exercer leurs fonctions et de fluidifier la circulation entre vie professionnelle et mandat local.

je le répète, la limitation du cumul des mandats dans le temps rendra ces garanties de plus en plus impérieuses. De même, je salue la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints,

le sénateur Darnaud, dont je partage l'analyse ; les pistes de réflexion vont dans le bon sens. Toutefois, s'il faut donner des garanties et renforcer les droits des élus, il ne s'agit nullement de les professionnaliser en revenant sur le principe de gratuité des fonctions électives. nécessaire d'étendre la formation des élus, le mécanisme de financement prévu à cet effet pourrait avoir des effets pervers et à rebours de l'objectif souhaité. Enfin, s'il faut limiter- c'est très

et alors que les discussions sont encore en cours avec les représentants des élus locaux, il est sans doute prématuré de se prononcer en faveur de mesures qui pourraient fortement évoluer dans les prochains mois. Cela alimenterait une insécurité juridique que dénoncent les élus locaux. Les élus communaux peuvent avoir confiance en nous, car, en privilégiant une réflexion globale et en étant force de proposition dans la concertation actuellement menée et dans les débats à venir cet automne, nous serons à même d'apporter des évolutions concrètes,

ainsi que l'illustrent les consultations, les rapports d'information publiés par les commissions et les délégations et les propositions de loi déposées par les sénateurs. Le texte que nous examinons cet après-midi constitue une nouvelle initiative sénatoriale, et l'on ne peut que s'en réjouir. En effet, face à l'insuffisance des garanties données aux élus locaux pour exercer leur mandat, cette proposition de loi offre des pistes intéressantes Toutefois, à titre personnel, je pense que l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux ne doit pas passer par la voie de la professionnalisation. Je le maintiens, être élu local n'est pas un métier, c'est un service rendu à la collectivité. L'élu local n'est pas rémunéré, il voit son engagement bénévole compensé, et cette compensation doit couvrir l'ensemble des frais liés au mandat. Un mandat, qu'il soit local ou national, découle d'une élection au suffrage universel

De façon plus générale, cette proposition de loi se heurte à un problème financier, car elle crée des contraintes nouvelles pour les collectivités territoriales, alors que le Sénat est toujours attentif à ne pas accroître inutilement leurs obligations. leurs obligations. L'impact financier d'un certain nombre de mesures proposées n'a malheureusement pas été pleinement mesuré. Par ailleurs, faisant suite aux propositions émises, par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, un projet de loi a été annoncé sur ce sujet pour la rentrée parlementaire. Des discussions sont en cours entre le Gouvernement et les représentants des élus locaux. monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants considère que ce texte arrive à contretemps et qu'il soulève des difficultés d'un point de vue financier. Il apportera sa contribution au débat, par le biais d'amendements déposés par ses membres, et il déterminera son vote à l'issue des discussions. La

Un certain nombre de choses ont été dites par les précédents orateurs, à commencer par Mathieu Darnaud ; je ne les répéterai évidemment pas, mais je veux exprimer la parfaite convergence

Bien évidemment, les insuffisances de ce que l'on a tendance à appeler le statut de l'élu et la difficulté à concilier l'exercice de fonctions électives avec la vie familiale et professionnelle se retrouvent aussi dans le discours de nos collègues. Plus que le statut de l'élu, ce sont bien évidemment les conditions de l'engagement préalable à l'élection, les conditions d'exercice

Ce travail très complet a sans doute servi de base au projet de loi en cours de rédaction. Le ministre Sébastien Lecornu exprimait il y a quelques minutes, à cette tribune,

utilement au débat qui s'engage sur les conditions d'exercice des mandats électifs. Je me réjouis de l'impatience exprimée par mes collègues à propos du futur texte gouvernemental, en cours de finalisation. J'en suis certain, nous pourrons l'enrichir ensemble. Je veux vous le dire, Pierre-Yves Collombat, ce

un moment qui n'est pas si simple du point de vue de la cohésion sociale et de la vie démocratique de notre pays. J'ai entendu deux appréciations du texte, de la part du ministre et de plusieurs intervenants : utilité et convergences.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat que nous allons engager est un débat du moment à en croire les annonces du Président de la République, qui parlait d'un « statut digne de ce nom », à en croire

En matière de dialogue entre l'État et les collectivités locales, on ne peut pas dire que l'année 2018 ait été caractérisée par la joie et la bonne humeur : contractualisation déséquilibrée, conférence nationale des territoires en échec,

le rôle indispensable joué par les bâtisseurs du quotidien que sont les élus locaux dans notre République, sans oublier, bien évidemment, la perspective des municipales de 2020 ... Monsieur le ministre, je partage votre

pourriez-vous demander à Mme Jacqueline Gourault de répondre à la question écrite que je lui ai posée en novembre 2018 et en janvier 2019 pour obtenir enfin une comptabilisation exacte, et par strate, des démissions d'élus.

d'avoir des informations pour avoir des informations, mais de savoir où ont lieu ces démissions. Cette question a toute son importance dans la définition du statut de l'élu. Cette vague de démissions et ces potentielles situations inédites que vous évoquez, monsieur le ministre, ont révélé publiquement le désenchantement qui touche les élus locaux.

du contexte d'exercice des mandats : technicisation, responsabilités croissantes, temps consacré aux mandats, exigence de nos concitoyens

L'ensemble de ces éléments a forcément un effet sur les politiques publiques choisies. Le statut de l'élu doit donc permettre d'ouvrir les fonctions électives à de nouveaux profils et d'éviter une représentation monolithique.

de pouvoirs exécutifs et les autres. Tous ces critères se superposent, ce qui amène nécessairement à prendre en compte cette complexité. Au risque de me répéter,

Pierre-Yves Collombat souligne que le statut de l'élu a pour but de « faciliter l'accession du plus grand nombre aux fonctions électives sans préjudice professionnel ou financier. Il doit permettre la représentation de la population dans toute sa diversité.

au titre de l'article 40, que nous chérissons tous -visant à reporter la suppression des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des syndicats.

! La proposition de loi pose une question fondamentale, celle de la persistance du mythe de l'amateurisme républicain.

depuis le 22 novembre 1906, depuis le débat sur l'augmentation de l'indemnité des parlementaires, la question de la professionnalisation revient comme un serpent de mer dans l'ensemble des discussions, sous les différentes Républiques. Ma collègue Élodie Lavignotte, auditionnée par le Sénat, soulignait que tous les textes parus depuis 1992 et la décentralisation conduisent, de fait, à une professionnalisation de certains mandats électifs locaux. pour des raisons à la fois historiques et liées à la tradition, l'exercice d'un mandat est toujours un entre-deux : entre métier et entre profession. Le principe de gratuité demeure le fondement de la légitimité de l'identité de l'élu, dans le même temps, toutes les dispositions viennent consacrer l'idée d'une professionnalisation. On peut chérir le mythe de l'amateurisme républicain et se rendre compte qu'il

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, si ce débat sur le statut de l'élu local arrive au bon moment, suite de la déclaration de politique générale du Premier ministre s'inspirant de ses expériences havraises, il arrive certainement au bon endroit, au Sénat, chambre des territoires. L'élu local est au coeur de la démocratie. À ce titre, il est désigné pour représenter nos concitoyens et conduire une collectivité, à savoir mettre en place les politiques publiques et les projets qui la font vivre. Premier interlocuteur des concitoyens, il est en contact direct et permanent avec eux, reprendre l'expression désormais célèbre et souvent citée de notre président Gérard Larcher. À cette fin, il exerce un mandat. Un principe historique préside à l'exercice de sa mission : la gratuité. Héritée de la pratique romaine, elle a été reprise dans les lois municipales de mars 1831 et confirmée par celle de 1884. C'est précisément cette gratuité qui fait la force de notre démocratie locale. Le mandat est libre, dénué d'intérêt pécuniaire. C'est un engagement citoyen au service de la collectivité, même si le principe de gratuité n'empêche pas une indemnisation, une compensation juste de cet engagement. Les travaux du Sénat et le rapport de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, intitulé, ainsi que de nombreux témoignages d'élus montrent que la conduite du mandat et l'engagement sont devenus très difficiles. Les facteurs sont identifiés et connus : multiplication des normes, manque de moyens, attentes fortes des citoyens, flou dans la répartition des compétences ... À un an des élections municipales,, en en partenariat avec l'Association des maires de France et le Cevipof, publiait ainsi une enquête sur le des élus locaux. La proposition de loi du sénateur Pierre-Yves Collombat et de plusieurs de nos collègues préconise la création d'un statut de l'élu communal et un ensemble de mesures lui garantissant un cadre sécurisé. Elle nous donne surtout l'occasion de débattre et de réfléchir sur un sujet très attendu par de nombreux élus et de trouver des solutions pour favoriser leur engagement dans un contexte ayant largement évolué ces derniers temps. Ce texte soulève toutefois quatre remarques de ma part. Tout d'abord, la création du statut de l'élu risque d'enfermer la personne dans un cadre strict et de figer le dispositif. C'est pourquoi j'ai souhaité déposer un amendement visant à poser les principes généraux des conditions d'exercice des mandats locaux. Ces dispositions, plus souples, permettent néanmoins de guider et d'éclairer les élus. Ensuite, la suppression de la gratuité du mandat remet en cause le sens historique de l'engagement volontaire et désintéressé des élus. Conférer une dimension pécuniaire revient à professionnaliser les élus locaux, en leur conférant les charges, les devoirs et les droits d'un salarié. L'élu local devient un salarié de la commune. Or je suis profondément opposée à ce changement de paradigme. C'est le sens de l'amendement que j'ai déposé, cosigné par plusieurs de mes collègues. Par ailleurs, l'impact financier de cette proposition de loi est fort pour les collectivités locales. Il me paraît à ce jour déraisonnable.

L'article 3 tend à renforcer ces obligations de formation et à instituer un fonds national pour la formation des élus locaux, qui serait alimenté par les communes. Toutefois, le mécanisme mis en place présente un double écueil d'ordre financier et politique la création d'un fonds national pour la formation des élus risque de conduire à nationaliser le financement de la formation des élus, ce qui reviendrait à brider l'autonomie des collectivités locales.

Cette proposition de loi est avant tout une occasion d'amorcer le sujet, dans la sérénité, pour que des solutions améliorant la vie pratique des maires soient définies et libèrent leur action au service de leurs concitoyens. La parole

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'heure où l'intercommunalité multiplie le nombre d'instances auxquelles participent les conseillers municipaux, à l'heure où la décentralisation a confié un nombre toujours croissant de responsabilités aux élus locaux, à l'heure où, d'élection en élection, l'âge moyen des maires augmente, à 'heure où le droit devient de plus en plus complexe à appliquer, nos élus locaux ont besoin, plus que jamais, d'un ensemble cohérent de dispositions régissant l'accès au mandat, l'exercice du mandat et la sortie du mandat. Je souhaite insister tout particulièrement sur la question de la fin de mandat, laquelle peut constituer un repoussoir au moment d'accepter de prendre des responsabilités municipales lorsqu'on a une carrière professionnelle devant soi. Chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de fluidifier la transition entre mandat local et vie professionnelle afin d'enrayer la crise des vocations électives et d'encourager les actifs à se porter candidats. Cette question de l'après-mandat devient une préoccupation essentielle pour tous les élus, au moment où notre démocratie tend à prendre la voie de la limitation du cumul des mandats dans le temps. Il existe donc une nécessité impérieuse de gommer les risques encourus en cas de non-réélection des élus locaux qui freinent le rajeunissement de la moyenne d'âge de nos maires. Le texte que nous examinons cet après-midi présente des pistes de réflexion intéressantes en vue d'offrir des garanties aux élus pour qu'ils puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions. En tout premier lieu, il a le mérite de reconnaître que l'investissement des élus, leur engagement, leurs responsabilités dépassent le cadre du bénévolat. Toutefois, permettra-t-il d'éviter une crise des vocations redoutée à l'occasion du scrutin municipal de 2020 ? Suffira-t-il à remonter le moral des maires que l'on dit découragés découragés et fatigués ? Je n'en suis pas sûr ... Les mesures proposées ne couvrent pas toutes les attentes des élus et leur impact financier pour les communes et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises, ne semble pas avoir été pleinement mesuré. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, un projet de loi a été annoncé pour l'automne sur ce sujet. Il sera présenté en conseil des ministres dès le mois prochain. Dans cette perspective, il apparaît primordial de trouver les solutions les plus adaptées et de dégager un consensus en poursuivant les concertations avec les représentants des élus locaux. Il sera également important de veiller à ne pas obérer davantage les capacités financières de nos collectivités. Aussi, dans ce calendrier, cette proposition de loi apparaît comme le préambule d'un débat nécessaire.

voté ce texte ... Il est temps d'avancer et d'aller au bout de cette démarche. Je tiens à remercier le groupe CRCE de cette belle initiative, qui va permettre d'ouvrir un débat fort utile, nécessaire, et qui, je l'espère, aboutira à des décisions concrètes pour les élus qui en attendent beaucoup. La

M. André Reichardt. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour, je voudrais rappeler que l'organisation territoriale française en un maillage communal est une particularité issue de la Révolution qui doit être sauvegardée du fait de ses nombreux bienfaits en termes de proximité avec les citoyens, de porosité aux problématiques qu'ils rencontrent et de lien social. Cependant, il aura fallu attendre la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux pour que le statut d'élu local connaisse une première concrétisation. Cette loi a été complétée par celle du 27 février 2002 et par celle du 31 mars 2015, laquelle comprenait une charte de l'élu local qui affirmait un certain nombre de principes s'apparentant déjà aux conditions d'une bonne gouvernance. Or, dans un contexte marqué par un déclin du civisme et par la complexification de l'exercice des mandats locaux, ces derniers principes doivent absolument s'accompagner des outils et des moyens suffisants pour faciliter l'exercice de ces mêmes mandats. Au regard du ras-le-bol de nombre d'élus, dont certains ont d'ores et déjà affiché leur volonté de ne pas se représenter en 2020, il est urgent d'instaurer un véritable statut de l'élu local qui permette aux citoyens qui le souhaitent de candidater aux prochaines élections municipales, avec la garantie de pouvoir articuler leur mandat électif avec une vie personnelle et professionnelle. cher collègue Collombat, si certaines pistes de réflexion proposées par les auteurs de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui sont intéressantes, voire même consensuelles, d'autres soulèvent des difficultés tant sur le plan juridique que financier. Je ne vais pas trop me répéter : il en va ainsi de l'article 3, qui propose d'étendre l'obligation de formation aux communes de 1 000 habitants et de créer un fonds national pour la formation des élus locaux, lequel serait abondé par les sommes non dépensées des formations complémentaires des communes de moins de 3 500 Dès lors, le financement des formations des petites communes serait transféré à un fonds national, faisant remonter les financements du niveau local au niveau national, pour ensuite redescendre au niveau local. Tout cela est un peu compliqué, pour ne pas dire cocasse. Si, sur un plan théorique, ce type de dispositif pourrait fonctionner à périmètre financier constant- je pense

actuellement réservé aux candidats des conseils municipaux des communes d'au moins 1 000 habitants, aux communes de plus de 500 habitants, appelle à la prudence. En effet, l'extension des garanties prévues pourrait peser, à des degrés divers, sur les finances des entreprises et des administrations qui emploient ces personnes. L'absence d'un salarié peut également être un facteur de désorganisation pour une entreprise, et ce à plus forte raison encore pour une petite entreprise artisanale ou commerciale.

pourrait peut-être conduire à une certaine « professionnalisation » de la fonction élective. Or un mandat local, tout comme un mandat national, ne constitue pas une activité professionnelle, mais un engagement civique au service de la collectivité. L'indemnité de fonction n'est donc pas une rémunération, mais une compensation

dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de certains syndicats mixtes. Malheureusement, l'amendement qui reprenait cette disposition, comme l'a souligné M. Kerrouche, a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, bien que parfois sévères vis-à-vis de l'action et de l'actualité politiques, les Français demeurent attachés à leurs communes, « cellules de base » de la démocratie, et à leurs maires. En tant que sénateurs représentant les collectivités territoriales et pour la plupart d'entre nous, exerçant ou ayant exercé des fonctions communales, nous savons mieux que quiconque l'importance des élus communaux, les difficultés du quotidien auxquelles ils sont confrontés, leur responsabilité pénale qui peut être engagée et, plus globalement, le manque d'attractivité du mandat- d'autres orateurs Il n'y a pas, selon moi, de mauvais moment pour en parler. Nous le savons, l'une des réponses à la crise sans précédent des « gilets jaunes » consiste à rebâtir une France plus unie et plus égalitaire à partir du terrain, partir des territoires, en s'appuyant notamment sur les élus locaux parfaitement au fait des problématiques de leur bassin de vie. Je rappelle d'ailleurs que leurs mises en garde à propos des effets des fractures territoriales sont restées lettre morte. On connaît la suite Au moment où le pays a plus que jamais besoin d'eux, nous ne pouvons plus continuer à compter uniquement sur leur bonne volonté et leur dévouement, car, à l'image d'autres serviteurs de l'intérêt général, comme les pompiers, les policiers ou la fonction publique hospitalière, beaucoup d'élus communaux sont las. Certains démissionnent, d'autres ne se représenteront pas. Les territoires les plus fragiles en seront les premières victimes. Dès lors, où et comment trouver des candidats disponibles, dévoués, désintéressés et compétents ? Certaines communes s'inquiètent déjà pour les prochaines élections Il faut donc les aider, car, comme l'a justement noté le rapporteur, améliorer les conditions d'exercice des mandats locaux constitue une ardente nécessité. C'est ce que propose de faire, bien qu'imparfaitement, la présente proposition de loi par la création d'un statut de l'élu communal assortie de diverses mesures. De façon générale, l'amélioration des conditions d'exercice des mandats communaux passe d'abord, à mon sens, par des moyens financiers accrus et un arrêt de la pression normative s'exerçant sur eux. Sans ressources suffisantes pour boucler leur budget, sans frein aux normes, l'exercice du mandat s'avérera toujours plus compliqué et éreintant, quelles que soient par ailleurs les mesures prises en faveur des élus.

envisageables pour mieux indemniser, former et protéger des élus locaux induisent une hausse des dépenses des collectivités territoriales, comme nous l'a rappelé notre collègue Reichardt. Les élus ont surtout besoin de stabilité. Les modifications permanentes du cadre juridique et institutionnel dans lequel ils évoluent- SCOT, intercommunalités, fiscalités, modes de scrutin et seuils -sont autant de facteurs de complexité et, souvent, de dépenses supplémentaires. S'y ajoute ce sentiment d'une administration de l'État toujours omniprésente, qui suggère ou dicte aux élus ce qu'ils ont à faire dans un pays pourtant largement décentralisé et alors même que le soutien des services de l'État aux collectivités s'est réduit. S'agissant précisément des mesures en faveur des élus, je ne crois pas opportun de supprimer le principe de gratuité pour ce qui concerne leurs fonctions, comme cela est proposé par la question du montant de leurs indemnités se pose, notamment dans les petites communes, de même que celle de leur fiscalité, vécue parfois comme complexe ou injuste. En outre, les élus communaux, en

qui nécessite de poursuivre la réflexion. Le Sénat a déjà beaucoup produit sur le sujet. Monsieur le

le président de la commission. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre intervention. Il y a certainement dans les propos que vous avez tenus les bases d'un travail en commun au service de nos collectivités territoriales. Vous le savez bien, le Sénat est ouvert à ce rappelé, vous avez été maire et président de conseil départemental. J'ai le souvenir d'avoir travaillé avec vous au sein du regroupement des cinq départements de Normandie, et je puis attester

des contrats aidés dont nos communes se servaient pour les cantines scolaires ou d'autres activités de service très utiles, le Gouvernement actuel est-il tout à fait décidé à lever un certain nombre d'obstacles à l'exercice des libertés locales

améliorer les capacités d'action des départements pour répondre, notamment, aux problèmes de développement économique qui leur sont soumis. Nous sommes prêts depuis longtemps. Vous avez sur la table la position du Sénat sur l'évolution nécessaire des dispositions de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.

mais sans précipitation, puisque la réflexion est sur la table depuis déjà plus d'un an sur certains sujets, voire plus sur d'autres. En effet, il nous semble que le fait de différer les modifications de la loi NOTRe serait une grave erreur par rapport aux attentes de nos collectivités.

Je ne suis pas sûr que nous comblerons le fossé qui les sépare en figeant la fonction de l'élu municipal dans un statut. Pour autant, je partage bien des dispositions figurant dans cette proposition de loi, laquelle s'inspire des recommandations formulées par notre délégation aux collectivités territoriales. Oui, il faut renforcer tout ce qui facilite l'exercice des fonctions électives ! En effet, il faut rompre avec la baisse d'attractivité des fonctions municipales, il faut veiller à la diversité des générations et des catégories socioprofessionnelles, au risque d'un repli sur une population d'élus déconnectés de la réalité de la société. Il faut également donner des moyens et une meilleure formation aux élus municipaux, afin qu'ils soient capables de peser face une technostructure de plus en plus spécialisée. En revanche, je ne pense pas que l'on se mette au service de la cité comme on entre dans un métier. Nous devons éviter de creuser un fossé entre des agents politiquement actifs sous statut et les autres citoyens, qui pourraient ainsi être encouragés dans leur passivité. Enfermer l'engagement municipal dans des règles rigides me semble aller à l'encontre de la promesse démocratique. Chaque citoyen est libre de participer à la vie démocratique ; c'est ainsi que notre pays a longtemps connu une remarquable vitalité de sa vie communale, qui fut un socle de notre République. Mes chers collègues, nous devons chercher à nourrir une plus grande convergence entre les différentes formes de participation des citoyens à la vie de la cité. Abolir le beau principe de la gratuité par la création d'un statut ne va pas dans le sens de la convergence entre démocratie directe et démocratie représentative. Telle est notamment la raison pour laquelle je réaffirme mon soutien à la position de M. le rapporteur. Je n'approuve pas l'abrogation de la gratuité des fonctions municipales.

C'est très vrai, car il s'agit d'une tâche enthousiasmante ! Pourtant, combien de fois ai-je perçu la lassitude des élus communaux ? Les motifs du découragement sont connus de tous : complexité des normes, réduction des moyens des communes et de leurs possibilités d'action en raison du transfert de compétences aux intercommunalités, risque juridique et pénal, insuffisance des mesures de compensation, problèmes de formation ou caractère insatisfaisant de la protection sociale, insuffisant soutien de l'État dans l'accompagnement des petites communes. Nous sommes tous d'accord : les conditions des mandats locaux doivent être améliorées. En outre, les moyens accordés doivent permettre d'aboutir à une réelle diversité sociologique et de genre. Comme le disait l'un de nos anciens collègues, toutes ces mesures auront un coût. Tel est le prix de la démocratie. Je partage donc le point de vue des auteurs de la proposition de loi concernant la nécessité d'aller vite.

lors de l'examen de chacun des grands textes traitant du statut des élus. Une telle suppression a toujours été repoussée, ce qui n'a pas empêché un certain nombre d'aménagements, certes insuffisants. Au demeurant, les termes du débat sont complexes. Si j'en crois certains chercheurs, l'exercice d'un mandat n'est ni un métier ni une profession, même s'il faut reconnaître que la fonction d'élu s'est fortement professionnalisée. L'élu rend service à la collectivité dès lors que son activité n'est pas rémunérée mais compensée, son engagement étant bénévole. La loi municipale ne dit pas autre chose ! Néanmoins, je note que, depuis longtemps, le renforcement des responsabilités des élus mérite un renforcement des compensations.

: je ne vais pas assez loin, ou trop loin, ce n'est pas le moment, ce n'est plus le moment, etc. La chose la plus réjouissante que j'ai entendue, c'est celle selon laquelle je serais à contretemps.

de citer, devant l'OIT : « Je crois que la crise que nous vivons peut conduire à la guerre et à la désagrégation de nos démocraties. J'en suis intimement convaincu. Je pense que tous ceux qui croient, sagement assis, confortablement repus, que ce sont des craintes qu'on agite se trompent. Ce sont les mêmes qui se sont réveillés avec des gens qui semblaient inéligibles ou sortis de l'Europe alors qu'ils pensaient que cela n'adviendrait jamais.

la fonction élective. Le code général des collectivités territoriales prévoit, pour ce qui concerne les maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux, que la fonction élective est gratuite. de ce texte nous proposent de revenir sur cette pétition de principe que je crois, pour ma part, essentielle. Mes chers collègues, la Révolution française

tout à fait enclins à poursuivre la discussion sur ce sujet.

le salarié ou l'agent fonctionnaire de la commune. Cette liberté, nous y tenons : tout mandat impératif est nul. Une fois que vous êtes maire, vous êtes libre. Cela ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi, cela veut dire que vous agissez en conscience. Enfin, je voudrais souligner que la dimension pratique de notre débat ne doit pas être perdue de vue. Ce matin, en commission des lois, sur l'initiative de notre rapporteur, M. Mathieu Darnaud, nous avons adopté un amendement

et mérite d'être mieux reconnu à travers le montant de l'indemnité. Plus la commune est petite, moins elle dispose de services techniques, ce qui contraint le maire et son adjoint aux travaux à être derrière les artisans quand on refait les huisseries de l'école

qui peuvent, le moment venu, ne pas renouveler son mandat, mais sa responsabilité est pleine et entière, et il ne saurait être qualifié de subordonné, même de ses électeurs.

de l'épanouissement des élus locaux, ni même pour favoriser leur engagement. Néanmoins, il paraît opportun d'intégrer à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, qui comporte déjà des dispositions relatives aux principes généraux

comme le soulignaient les auteurs du rapport de 2018 sur l'exercice des mandats locaux. Au surplus, la proposition de loi comporte de nombreuses mesures incrémentielles visant à améliorer les conditions d'exercice de ces mandats, mais ne se place pas dans la perspective d'un travail d'ensemble, codifié et plus profond. Pour ces raisons, le présent amendement tend à substituer aux dispositions créant un statut de l'élu d'autres dispositions, plaçant dispositions, plaçant les principes généraux d'exercice des mandats locaux dans le cadre plus général des dispositions du code général des collectivités territoriales. Le renvoi aux « principes généraux permet également de prévenir tout risque juridique lié à la présence de dispositions s'appliquant aux élus locaux dans d'autres codes, notamment le code du travail et le code électoral.

le code général des collectivités territoriales. Dès lors, afin de renforcer la clarté, l'intelligibilité et la concision de la norme, il paraît opportun de privilégier une rédaction plus brève de cet article.

même pour la troisième entrée : « situation de fait, position, par rapport à la société, aux institutions, etc. : le statut de la femme, du livre ». Pourquoi pas de l'élu territorial

en plus d'être une tradition, relève d'une certaine vision de l'engagement démocratique local : l'indemnisation ne se veut pas la contrepartie d'un service de type professionnel ni la rémunération d'un travail fourni.

sauf à vouloir faire référence au statut de la fonction publique : ce n'est tout de même pas le modèle que nous voulons prendre pour définir l'ensemble des textes et des règles qui seront applicables aux élus locaux

créer d'abcès de fixation sur l'usage d'un mot qui n'a pas à proprement parler de définition juridique : le mot « statut » n'a pas de statut juridique

Concilier vie professionnelle et exercice d'un mandat électif est l'une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les élus locaux.

pour l'exercice d'un mandat électif. Par ailleurs, cet article prévoit d'augmenter le volume du crédit d'heures. Le volume actuel- jusqu'à 140 heures au maximum par trimestre selon la taille des communes -est jugé nettement insuffisant par les maires. Nombre d'entre eux sont contraints de mettre entre parenthèses leur carrière professionnelle, de passer à temps partiel, avec toutes les conséquences que cela entraîne à la fin du mandat. Mais tous ne le peuvent pas ou ne le souhaitent pas. Il s'agit, là aussi, de favoriser l'exercice des responsabilités électives.

aux candidats aux élections municipales et aux conseillers municipaux, lorsqu'ils sont salariés, afin de leur permettre de participer à la campagne électorale et à l'administration de leur commune.

dans l'articulation de l'article 2. Il vise en effet à harmoniser la rédaction proposée avec celle de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, qui établit une tranche de population allant de 500 à 1 499 habitants. Or la formulation actuelle reviendrait à fixer un seuil à 501 habitants. Afin de ne pas multiplier les seuils et de ne pas complexifier inutilement le droit des collectivités territoriales, il paraît préférable d'unifier les rédactions.

pour présenter l'amendement n° 62. Outre que de telles duplications ne produiraient aucun effet juridique, elles nuiraient à la lisibilité du droit et risqueraient de provoquer des incohérences dans le cas où l'un ou l'autre des deux codes viendrait à être modifié à l'avenir. Par ailleurs, on comprendrait mal que ne soient reprises dans le code du travail que les dispositions relatives aux conseillers municipaux et non celles, de même objet, qui concernent les autres élus locaux.

à M. le rapporteur. Les conseillers communautaires des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ont la possibilité de bénéficier de crédits d'heures et d'autorisations d'absence pour leur permettre de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur mandat. Une telle possibilité n'est pas prévue pour les conseillers communautaires des communautés de communes. de communes. Au vu des compétences croissantes de cette catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette exception ne semble pas justifiée. Cet amendement vise donc à permettre aux conseillers des communautés de communes de bénéficier de crédits d'heures et d'autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les autres conseillers communautaires.

Je rappelle que le décret de juin 2016 relatif à la cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnités de fonctions pour le financement du droit individuel à la formation des titulaires de mandats locaux prévoit une cotisation des élus locaux bénéficiant d'indemnités de fonctions pour le financement de ce droit, fixée à 1 % du montant brut annuel de ces indemnités. Depuis 2016, 14 millions d'euros sont prélevés à ce titre chaque année sur les indemnités des élus locaux, soit un total de 42 millions d'euros à la fin de l'année 2018. Néanmoins, seuls 2 millions d'euros ont été véritablement utilisés par les élus locaux au titre du DIF en 2017 et en 2018. On peut donc légitimement s'interroger sur la pertinence du montant des cotisations obligatoires acquittées par les élus locaux pour financer un fonds consacré à leur formation.

y apporter des modifications susceptibles de le rendre plus efficient et de consolider ainsi le droit à la formation de nos élus. La parole

La démocratie représentative implique que chaque citoyen puisse, à l'occasion d'élections libres, être élu et avoir l'honneur de représenter la Nation. Les décideurs locaux présentent une diversité sociologique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Cet idéal démocratique ne doit cependant pas occulter le fait que la conduite des affaires publiques nécessite aujourd'hui de larges compétences. Le mandat local s'est épaissi, dans un environnement juridique et technique plus complexe. Désormais, l'élu local doit disposer de connaissances suffisantes pour prendre les bonnes décisions. S'il exerçait initialement une fonction représentative, il est aujourd'hui devenu un véritable gestionnaire. Dans cette optique, le droit à la formation des élus apparaît comme une véritable condition du bon exercice du mandat. J'irai même plus loin, en affirmant que la préservation de la capacité de décision autonome des élus locaux est une condition même de la libre administration des collectivités territoriales. Depuis 2012, j'ai pu prendre la mesure du chemin accompli en matière de droit à la formation des élus locaux.

ces difficultés ont été confirmées. Ainsi, près de 97 % des répondants indiquent n'avoir « jamais bénéficié d'un congé pour suivre une formation ». Près de 70 % des répondants indiquent n'avoir bénéficié « d'aucune prise en charge de frais afférents à une formation » et 99 d'aucune compensation par la collectivité des pertes de revenus subies » dans ce cadre. Je suis donc naturellement favorable à la première mesure inscrite à cet article, à savoir l'obligation de formation pour les élus des petites communes. Mais encore faut-il que les élus soient incités à suivre des

c'est avoir la confiance de ses concitoyens, cette confiance reposant sur la capacité à maîtriser les dossiers soumis aux assemblées locales. Or, la légitimité du suffrage universel n'induit pas automatiquement la connaissance.

les nombreux élus des toutes petites communes, pourtant souvent seuls face à leurs responsabilités. Dois-je rappeler le contexte de complexification de l'action publique locale et la nécessité de posséder des compétences pointues, quelle que soit la taille de la commune

en envisageant l'extension de cette obligation à l'ensemble des communes, en tout cas pour les élus ayant reçu une délégation. Cela impliquerait évidemment, je le reconnais, de régler les questions du financement et de la revalorisation des dotations.

par la Caisse des dépôts et consignations. Il est proposé que cette information ne soit pas réservée aux seules commissions des finances des deux assemblées, mais qu'elle soit adressée à l'Assemblée nationale et au Sénat dans leur globalité.

Cet amendement tend à prévoir que le Comité des finances locales décide chaque année du taux de la cotisation obligatoire en fonction du niveau de consommation du fonds.

? L'amendement vise à porter le seuil à compter duquel les communes doivent obligatoirement organiser une formation pour les membres du conseil municipal ayant reçu délégation de 1 000 à 1 500 habitants. Or c'est justement dans les petites communes,

Cet amendement vise à ce que chaque assemblée locale définisse un plan pluriannuel de formation pour la durée du mandat.

du mandat des membres du conseil municipal est inférieure à six ans. Il est donc proposé de préciser que ce plan de formation est établi « pour la durée restant à courir des mandats des conseillers municipaux

soulève un certain nombre de problèmes techniques et juridiques. Il tend, par la péréquation, à nationaliser le financement de la formation des élus, ce qui nous paraît contraire au principe de libre administration des collectivités.

aux crédits qu'elles inscrivent pour la formation de leurs élus. En outre, il existe déjà une aide visant à permettre aux plus petites communes de financer leurs actions de formation : il s'agit de la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux. L'éligibilité à cette dotation pourrait

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous rappelle que la présente proposition de loi a été inscrite par la conférence des présidents dans le cadre de l'ordre du jour réservé au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, c'est-à-dire pour une durée de quatre heures. Les quatre heures quatre heures étant écoulées, je me vois dans l'obligation d'interrompre l'examen de ce texte. Il reviendra à la conférence des présidents d'inscrire la suite de cette proposition de loi, ainsi que la proposition de loi suivante, dont nous n'avons pas pu entamer l'examen, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.